La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 13 avril 2023 a été publié sur le site internet du sénat.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'inclusion de l'hydrogène nucléaire aux côtés de l'hydrogène renouvelable dans les textes européens en cours de négociation, qu'il s'agisse de la révision de la directive sur les énergies renouvelables ou du règlement pour une industrie à zéro émission nette,

aussi contraire à notre souveraineté énergétique, car l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consacre le droit des États membres de choisir entre ces différentes sources d'énergie. C'est enfin mal avisé au regard de la compétition internationale : l'Europe ergote sur la définition de l'hydrogène, alors que les États-Unis, dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation (), accordent une remise fiscale allant jusqu'à 3 euros par kilogramme sur l'hydrogène décarboné, quelle que soit son origine. Que de moyens gâchés, que de temps perdu, que d'opportunités manquées, ici, en Europe ! Or l'hydrogène est un vecteur de premier plan pour réussir notre transition énergétique. énergétique. Il permet, d'une part, de décarboner certains secteurs, en particulier l'industrie et les transports, d'autre part, de stocker l'électricité. Cette capacité de stockage est essentielle pour promouvoir la mobilité propre, en complément des batteries électriques, ainsi que les énergies renouvelables, qui pèchent toujours par leur intermittence. Dans ce contexte, la commission des affaires économiques du Sénat s'est mobilisée en faveur de l'hydrogène bien avant le Gouvernement- et bien souvent contre lui. Dans la loi Énergie-climat de 2019, nous avions fixé un objectif de 20 % à 40 % d'hydrogène décarboné d'ici à 2030 du développement de ses usages dans l'industrie, l'énergie et la mobilité. Dans notre plan de relance Énergie, publié en juin 2020, en pleine crise de la covid-19, nous avons appelé à « révéler le potentiel de l'hydrogène

Plus récemment, dans notre rapport sur l'énergie nucléaire et l'hydrogène bas-carbone, publié en juillet 2022, nous avons plaidé pour « saisir l'occasion de la relance du nucléaire pour favoriser une production massive d'hydrogène bas-carbone Cela nous a conduits à consolider la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables de mars dernier : d'une part, nous avons imposé un bilan carbone à tous les projets d'hydrogène soutenus par appels d'offres, afin de favoriser les projets les moins émissifs et les plus circulaires

enfin adopté plusieurs mesures de simplification en instituant un guichet unique et en consolidant les opérations d'autoconsommation et les plateformes industrielles.

texte est le fruit du compromis issu de la commission mixte paritaire sur le projet de loi Énergie-climat de 2019. Convaincus de la nécessité d'inverser la hiérarchie des normes en matière énergétique, nous avions souhaité établir la primauté de cette loi quinquennale sur les documents de planification réglementaires. Face aux changements climatiques qui posent aussi un défi démocratique, nous avions voulu affirmer la préséance du législateur sur le pouvoir réglementaire, celle de la politique sur la technique.

Dans notre résolution sur le paquet Ajustement à l'objectif 55 d'avril 2022, nous avons plaidé en faveur de la même vigilance. L'hydrogène bas-carbone ne doit pas être pénalisé par la directive sur la taxation de l'énergie ni être exclu de la directive sur les énergies renouvelables

recharge. L'hydrogène doit être activement soutenu, tant dans les processus de l'industrie que dans les modes de transport. Pour y parvenir, une stratégie claire, une gouvernance solide, des financements pérennes et une réglementation idoine

pouvez-vous nous indiquer quelles dispositions sur l'hydrogène nucléaire ou renouvelable comportera la prochaine loi quinquennale de programmation sur l'énergie et le climat ? Pouvez-vous également nous préciser comment la France entend défendre l'hydrogène nucléaire dans le cadre du paquet Ajustement à l'objectif 55 ?

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs,

Pour autant, le mix énergétique de demain sera plus diversifié que celui d'aujourd'hui. L'électricité, nous le souhaitons, deviendra majoritaire juste

Ces usages sont stratégiques, car ils concernent les industries de base. Garantir l'accès à de l'hydrogène bas-carbone- ce dernier terme est important -est un choix de souveraineté industrielle qui permettra de maintenir sur notre territoire des industries lourdes, qui ne peuvent se décarboner sans hydrogène.

de l'hydrogène sur le territoire est certes un défi, mais cela présente des avantages importants : devenir souverain en maîtrisant cette technologie et en faire un véritable facteur d'attractivité pour les investisseurs internationaux.

Nous pouvons nous réjouir qu'une stratégie française de l'hydrogène vert se dessine enfin, stimulée notamment par le paquet européen Ajustement à l'objectif 55. Les objectifs fixés sont clairs et ambitieux : remplacer progressivement l'hydrogène gris, qui représente actuellement plus de 90 % de la production, et parvenir à l'installation de 6,5 gigawatts d'électrolyse en 2030, soit la production de 600 kilotonnes par an d'hydrogène décarboné. Plusieurs sites de production commencent à se déployer sur le territoire. À cet effet, de nombreuses aides sont mises en place : soutien des investissements déterminants pour la construction d'une véritable filière d'hydrogène vert à hauteur de 7 milliards d'euros dans le cadre de France 2030, aides du fonds européen de développement régional, dispositifs de soutien aux démonstrateurs ainsi qu'aux écosystèmes territoriaux l'Ademe et les programmes d'investissements d'avenir, mécanismes de soutien réservés aux grands projets d'intérêt européen Tout cela nourrit une dynamique plutôt enthousiasmante pour la transition énergétique de notre économie et de nos territoires, comme je le constate dans ma région. Néanmoins, un défi majeur demeure : celui du développement des usages, que ce soit dans l'industrie ou dans la mobilité. En effet, l'acquisition d'un bus ou d'un camion à hydrogène reste extrêmement coûteuse pour les entreprises et les collectivités locales. Le plan rétrofit et le plan de soutien à la décarbonation des cinquante sites les plus polluants ne contiennent que quelques mesures timides en matière d'usage d'hydrogène vert. Il faut donc proposer de véritables incitations, notamment financières, comme nous l'avons fait pour l'électricité ou les biocarburants. Seule une augmentation de la demande permettra de faire baisser le prix de production. Monsieur le ministre, quelle politique d'incitation le Gouvernement compte-t-il mettre en oeuvre pour le développement de la production d'hydrogène vert, qui s'accompagne d'une massification de son usage dans tous les secteurs de l'économie ?

Menonville. Monsieur le ministre, développer l'hydrogène au sein de notre mix énergétique, c'est allier la transition énergétique avec une politique industrielle efficace et ambitieuse. Alors que la France a fait le choix de la relance de sa filière électronucléaire, elle ambitionne également de développer une filière hydrogène décarbonée s'appuyant tant sur le développement des énergies renouvelables que sur notre filière nucléaire. C'est la garantie de notre souveraineté et de notre indépendance énergétiques, alors même que d'autres pays européens s'orientent plutôt vers de l'hydrogène issu d'énergies exclusivement renouvelables renouvelables et vers des importations. La situation géopolitique actuelle nous appelle à plus d'autonomie aux niveaux français et européen.

Cela sera-t-il suffisant pour faciliter la production d'hydrogène bas-carbone ? À quelques semaines de l'examen du projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat, pouvez-vous nous préciser quelle place y tiendra l'hydrogène ? Quelle articulation comptez-vous bâtir entre les énergies renouvelables, la filière électronucléaire et l'hydrogène ?

M. Daniel Salmon. Monsieur le ministre, à la différence de l'électricité, l'hydrogène est une énergie de stock et non une énergie de flux. C'est là tout son intérêt : il peut être associé à des énergies intermittentes ou variables, comme le solaire et l'éolien. Il a donc toute sa place dans notre mix énergétique.

Alors que le projet de pipeline H2Med entre la péninsule ibérique et la France a été lancé, la politique française s'appuiera-t-elle majoritairement sur ces importations ? Envisagez-vous le développement de l'hydrogène une production locale avec des énergies renouvelables ? Vous avez donné quelques

? La parole est à M. Frédéric Marchand. S'appuyer sur nos laboratoires de recherche et sur nos industriels à la pointe de l'innovation, créer une filière compétitive d'hydrogène renouvelable et bas-carbone et devenir l'un des leaders mondiaux de l'hydrogène décarboné par électrolyse : telle est la feuille de route de notre pays pour offrir à l'hydrogène un futur prometteur dans notre mix énergétique, il est indispensable de lever certains freins, en améliorant le rendement des procédés de production, en optimisant le stockage à haute pression ou encore en favorisant les investissements, de réduire autant que possible le risque industriel. Il semble donc incontournable de mettre en place des politiques publiques visant à encourager le déploiement et la baisse de coûts de certaines technologies. L'Union européenne et ses États membres ont récemment réaffirmé leur intention de mettre en oeuvre des contrats pour la différence,

admettait surtout que la voiture individuelle à l'hydrogène restait un mythe, faute d'attrait économique. Après avoir tranché les questions de production, comment le Gouvernement prévoit-il d'accompagner la démocratisation

Aujourd'hui, la stratégie nationale hydrogène se décline en trois objectifs issus du plan d'investissement France 2030 : installer suffisamment d'électrolyseurs pour décarboner l'économie, développer les mobilités propres et construire une filière industrielle en créant 50 000 à 150 000 emplois. Monsieur le ministre, se tourner vers le futur ne doit pas empêcher d'apprendre des erreurs du passé,

mais il ne faut pas se voiler la face : les États-Unis, qui subventionnent massivement l'hydrogène décarboné, sont pour l'instant bien plus attractifs que nous. Si, demain, tel ou tel industriel privé décide de fermer des sites français au motif qu'il serait plus rentable de s'installer outre-Atlantique, de quelle maîtrise la France disposera-t-elle ? Concrètement, nous devrons réinvestir des milliards et des milliards d'euros sous peine de voir s'effondrer la filière et prendre une nouvelle fois du retard.

Ambitieux pour certains, utopique pour d'autres, cet objectif passera nécessairement par la multiplication de nos capacités d'importation d'énergie d'origine renouvelable. Dans cette perspective, l'Union européenne a d'ores et déjà signé des protocoles d'accord avec nombre de pays, notamment africains, afin de bénéficier de leurs capacités de production d'énergies renouvelables. Toutefois, un certain nombre d'observateurs alertent dès à présent quant aux limites d'un fort recours à l'importation. En effet, les pays exportateurs d'énergies renouvelables devront puiser dans leurs réseaux nationaux pour fournir l'énergie nécessaire à l'Union européenne, au détriment des populations locales. L'exemple de la Namibie est particulièrement éloquent. En 2022, seuls 56 % des Namibiens avaient accès à l'électricité. Pourtant, leur pays se dit prêt à exporter en masse sa production d'énergies renouvelables vers les États européens. L'accord trouvé avec l'Union européenne est symbolique de cette dynamique dramatique. Afin de développer l'hydrogène vert,

Notre transition énergétique sera mondiale ou ne sera pas. Il est de notre responsabilité de la concevoir à l'échelle mondiale. Monsieur le ministre, ferons-nous le pari de l'hydrogène vert s'il implique une dépendance toujours plus grande d'autres pays aux énergies fossiles ?

permettant d'éviter l'émission de 6 millions de tonnes de CO2 par an. On ne peut qu'approuver un tel objectif. L'hydrogène dit vert ou décarboné obtenu par électrolyse est non seulement une manne pour le développement des énergies renouvelables, mais aussi un vecteur incontournable pour la décarbonation de secteurs comme l'industrie lourde, les mobilités routières intensives ou les transports maritimes et aériens. Toutefois, je tiens à soulever quelques questions concernant l'amont de sa production. L'hydrogène par électrolyse mobilise la ressource en eau. Ainsi, la production d'un million de tonnes d'hydrogène renouvelable et bas-carbone nécessiterait entre 10 millions et 20 millions de mètres cubes d'eau.

de nouvelles synergies pour la réutilisation des eaux usées industrielles, le développement des technologies de désalinisation partielle ou encore l'utilisation d'eau marine dans l'industrie ? Je souhaiterais connaître votre avis sur ces différentes pistes. L'autonomie minière est également un enjeu majeur. la filière hydrogène n'échappe pas aux besoins en métaux critiques, tels que l'iridium et le platine. Alors que la production de platinoïdes est concentrée dans quelques pays, dont certains sont fragiles sur le plan géopolitique, et que la dynamique autour de l'hydrogène est très importante, en Europe comme dans d'autres régions du monde, comment sécuriser l'approvisionnement de la filière hydrogène pour les prochaines décennies ? Enfin, sur les

l'industrie du décolletage, très présente dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, que vous connaissez, est menacée par la fin des moteurs thermiques d'ici à 2035 : elle voit dans ces nouvelles technologies une importante vous-même : considérer l'hydrogène comme une solution miracle appelée à remplacer les autres formes d'énergie reviendrait à se méprendre. Son usage ne peut s'inscrire qu'en complémentarité avec les énergies renouvelables telles que le photovoltaïque, l'hydroélectricité et l'éolien, lesquelles devront nécessairement monter en puissance pour que la France puisse produire suffisamment d'hydrogène. même en accélérant notre production d'énergie renouvelable, la France et plus largement l'Union européenne ont nettement moins de potentiel de production renouvelable que des pays situés sur d'autres continents. Il est donc essentiel que l'hydrogène produit grâce à l'énergie nucléaire, également appelé hydrogène rose, puisse être considéré comme renouvelable.

Redon-Sarrazy. Monsieur le ministre, nous dressons un même constat quant à l'utilité de l'hydrogène pour accélérer la transition énergétique. L'hydrogène peut effectivement contribuer au basculement progressif vers les énergies renouvelables, mais encore faut-il s'entendre sur son mode de production.

provient à 69 % du gaz naturel et à 27 % du charbon, le reste étant fourni par l'électrolyse de l'eau et d'autres solutions plus vertueuses. Sa production n'a donc entraîné aucune décarbonation des économies. L'hydrogène doit évoluer vers un mode de production décarboné, idéalement en passant par une source d'électricité renouvelable. La voie offerte par l'électrolyse est intéressante à plusieurs égards. Elle utilise l'énergie électrique pour récupérer l'hydrogène présent dans l'eau. De plus, en couplant un électrolyseur à une source décarbonée d'électricité, l'on obtient de l'hydrogène vert, qui n'émet pas de CO2.

Par ailleurs, l'hydrogène électrolytique suppose des infrastructures complexes, non seulement de production, mais aussi de transport et de distribution, et des capacités de stockage. On estime que le déploiement de telles infrastructures ne pourrait se faire avant le milieu de la décennie. Dans l'attente, on persistera à produire de l'hydrogène carboné, à moins que l'État n'engage une stratégie clairement définie en la matière. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous détailler le calendrier que l'État entend suivre pour développer une filière de production d'hydrogène vert ?

la France dispose d'atouts technologiques et d'une politique offensive d'accompagnement financier des projets, au travers du plan hydrogène 2030, et c'est réellement une très bonne chose. Pour peu qu'il soit vert, c'est-à-dire produit à partir d'énergies renouvelables, l'hydrogène peut décarboner trois grands secteurs d'activité : les mobilités, l'industrie et le chauffage des bâtiments. Les transports, lourds et en commun, bénéficieront de cette technologie à moyen terme, tout comme l'industrie de fabrication d'acier et de ciment, actuellement très polluante. Quant aux bâtiments, ils pourraient profiter de la mise sur le marché des premières chaudières faisant appel à la technologie de la condensation de gaz.

blanc ? Ce concept est très récent, car l'hydrogène a longtemps été considéré comme un gaz n'existant pas naturellement sous sa forme moléculaire dans le sous-sol. Or ce postulat vient d'être contredit par de récentes expérimentations menées au Mali, aux États-Unis, en Australie ainsi qu'en Chine. Les réserves mondiales étant considérables et le prix d'extraction très inférieur à celui de la fabrication, des demandes d'autorisation de recherche provenant de sociétés françaises ont été formulées. L'État français envisage-t-il d'y répondre favorablement ? La parole est à M. le ministre

évidemment préjuger de leur instruction : l'État doit déterminer, selon le code minier, l'ampleur du potentiel de gisement, les fondamentaux économiques et les bénéfices environnementaux réels. Nous nous attacherons bien sûr à remplir ces trois conditions. Mes Mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer, dans la tribune d'honneur, une délégation de sénateurs polonais, conduite par M. Aleksander Pociej, président du groupe d'amitié Pologne-France. Elle est accompagnée par notre collègue Mme Valérie Boyer, présidente du groupe d'amitié France-Pologne. Cette visite d'étude permettra de renforcer la coopération franco-polonaise dans le contexte particulier du conflit en Ukraine. Ses travaux concerneront le domaine de la défense, mais aussi le secteur agricole et la coopération en matière scientifique.

Mes chers collègues, à la veille du 3 mai, qui est une fête nationale en Pologne, célébrant la Constitution du 3 mai 1791, je souhaite, en votre nom à tous, à nos homologues du Sénat polonais, la plus cordiale bienvenue ainsi qu'un excellent et fructueux séjour.

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire concrètement comment le Gouvernement va s'assurer que ces entreprises, issues de la filière française de l'électrolyse pour l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, trouveront des débouchés suffisants d'ici à 2030 qui leur permettront de se consolider, de devenir des fleurons industriels durables pour notre pays bénéficier sur le long terme de notre position de nation pionnière dans ce domaine

au développement de la mobilité professionnelle- des véhicules utilitaires légers aux camions, des bennes à ordures aux autobus -et de la mise en place d'infrastructures de recharge hydrogène maillant l'ensemble du territoire national. ne doivent être ni retardés ni négligés dans la révision de la stratégie nationale. Alors que la France a la chance de compter deux constructeurs automobiles ayant mis au point des véhicules utilitaires légers à hydrogène, il serait véritablement regrettable de ne pas potentialiser cette avance technologique au moment où les zones à faibles émissions (ZFE) vont être mises en oeuvre.

comme un moyen de décarbonation de l'énergie de filières industrielles particulières, que vous avez d'ailleurs évoquées, monsieur le ministre. Pour autant, on parle peu des solutions que l'hydrogène devra apporter pour permettre le bon fonctionnement de l'ensemble du parc national de production d'électricité. Plus précisément,

Dit autrement, plus la part d'énergies renouvelables dans le mix énergétique sera importante, plus nous aurons besoin de faire appel à la fonction particulière de stockage de l'hydrogène. La compétitivité des énergies renouvelables sera aussi fonction de la contribution de l'hydrogène à la flexibilité et à l'équilibre du réseau en situation de moindre disponibilité des énergies renouvelables. Toutefois, cette contribution à la flexibilité du réseau nécessite des infrastructures de stockage et de transport d'hydrogène importantes. Pour y parvenir, il est indispensable d'intégrer au mix énergétique et au réseau d'énergie électrique national un système hydrogène composé d'électrolyseurs, de stockages d'hydrogène, de points d'avitaillement, de centrales thermiques à hydrogène, de réseaux de transport, voire d'interconnexions avec les pays limitrophes. En définitive, la nature et l'ampleur du système hydrogène qui serait intégré à la régulation du réseau électrique national conduiraient à plus ou moins de flexibilité. Un tel choix politique- c'en est un ! -aura des conséquences sur les niveaux d'énergies renouvelables dans le mix et donc sur la PPE. sur la PPE. Monsieur le ministre, quelle est la doctrine du Gouvernement en matière de gestion de la flexibilité du futur réseau électrique national ? Quel type de système hydrogène entendez-vous développer en matière de flexibilité ? Où en êtes-vous de la planification des investissements nécessaires ? Comment et sur quels acteurs les coûts de ces investissements seront-ils répercutés ? La parole

Mme Béatrice Gosselin. Mes chers collègues, à condition qu'il soit produit par des moyens ne conduisant pas à des émissions significatives de carbone, l'hydrogène présente l'intérêt d'être, d'une part, un vecteur énergétique de choix pour certaines industries ou pour la mobilité lourde et, d'autre part, un outil de flexibilité du mix électrique qui aide à décarboner des secteurs difficiles à électrifier. Comme énergie, l'hydrogène bas-carbone est applicable au secteur de la mobilité- transport collectif de personnes et transport de marchandises -, là où les solutions à base de batterie sont plus difficiles à mettre en oeuvre ou soulèvent des enjeux majeurs. Utilisé dans une pile à combustible, il présente l'avantage de ne rejeter que de l'eau, ce qui permet d'éliminer les émissions de particules, de soufre, d'oxyde d'azote et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air.

Pour autant, c'est bien l'électrolyse de l'eau qui représente l'avenir du développement de la filière hydrogène. Le projet en Vendée, plateforme en mer raccordée à une éolienne flottante, s'avère être une perspective intéressante pour la production d'hydrogène renouvelable. En effet, après désalinisation de l'eau de mer, l'hydrogène sera produit par électrolyse et acheminé sur terre un réseau de pipelines. Mais le défi immédiat, pour accompagner la production par électrolyse d'hydrogène propre, consiste à assurer un approvisionnement suffisant en électricité décarbonée. pour atteindre les objectifs de décarbonation fixés par la Commission européenne en 2030, l'hydrogène bas-carbone produit à partir d'électricité nucléaire sera-t-il reconnu comme indispensable, à l'instar de l'hydrogène renouvelable ? La parole

Ce complexe utilise près de 75 000 tonnes d'hydrogène par an produit, pour l'instant, à partir de gaz, ce qui est très émetteur de CO2. Pour passer à l'hydrogène vert, il faudrait un électrolyseur d'une capacité de 500 mégawatts, sachant que la plateforme chimique pourrait utiliser la chaleur fatale de ce dernier. Cet avantage en matière d'optimisation énergétique pourrait conduire à une augmentation de 100 mégawatts de capacité pour fournir de l'hydrogène décarboné pour le transport, par exemple. Mais avec la forte variation du coût du gaz en Europe, nettement plus cher que le gaz américain ou russe, ces entreprises ont dû réduire leur production, faute de pouvoir exporter. Butachimie, par exemple, ne tourne plus qu'à 30 % de sa capacité. Dans ce modèle économique intégré, si l'une de ces entreprises venait à cesser son activité, cela entraînerait de sérieuses difficultés pour les deux autres. Le Gouvernement veut passer à l'hydrogène vert, produit par électrolyse. Toutefois, avec l'explosion des prix de l'énergie, cela semble très mal engagé. Les aides plafonnées à 4 millions d'euros ne sont pas suffisantes pour des entreprises de cette taille, car une différence de 1 euro sur le prix du kilogramme d'hydrogène représente une perte de 75 millions d'euros. Il faut absolument revoir notre modèle de soutien à cette industrie, afin de pérenniser les installations actuelles et leur donner de la visibilité. À défaut, sur ce seul site,

Monsieur le ministre, que compte faire le Gouvernement pour soutenir cette industrie et les investissements qu'elle va devoir engager pour passer à l'hydrogène vert ? Quelles actions vont être mises en oeuvre pour soutenir ce complexe chimique, afin d'empêcher un nouveau désastre économique ? La parole

Merci

pourtant, depuis la découverte fortuite, voilà presque dix ans, d'un puits d'hydrogène presque pur au Mali, qu'il existe de nombreuses sources d'hydrogène naturel un peu partout dans le monde. Aussi, l'hydrogène constitue une source d'énergie primaire à extraire du sous-sol.

des poches d'hydrogène qui intéressent beaucoup les sociétés de prospection. L'une d'entre elles a déposé une demande de prospection exclusive sur un périmètre de 226 kilomètres carrés dans les Pyrénées-Atlantiques. Si le projet aboutit, un chantier de production d'hydrogène comme source d'énergie primaire décarbonée et disponible en permanence sera lancé avec un coût de production de moins de 1 euro le La France ne peut ignorer cet énorme potentiel ! Je souhaite donc savoir si le Gouvernement compte accompagner le mouvement en encourageant et en encadrant les opérations de prospection et d'exploitation, qui vont se multiplier, notamment dans les Pyrénées-Orientales, puisque la présence d'hydrogène et de failles en profondeur a été confirmée dans l'ensemble du massif pyrénéen.

la production de 1 million de tonnes d'hydrogène sur notre territoire, essentiellement par vaporeformage du méthane, engendre plus de 11 millions de tonnes de dioxyde de carbone. L'enjeu, bien identifié, est donc de parvenir à des modes de production neutres en CO2. Tel est le deuxième défi auquel nous sommes confrontés : comment concilier les promesses intrinsèques de ce vecteur énergétique avec des réalités économiques et écologiques qui lui sont aujourd'hui encore assez défavorables ? Comme ? Comme pour toute filière novatrice, les coûts de production de l'hydrogène bas-carbone, essentiellement par électrolyse de l'eau, sont encore élevés- jusqu'à 8 euros le kilogramme contre environ 2 euros pour l'hydrogène gris. La marche est haute et l'équilibre ne pourra être atteint sans aides publiques importantes à l'investissement, surtout si l'on veut doubler le volume produit d'ici à 2028 à hauteur de 20 % de la production globale.

point crucial pour la rentabilité de la filière hydrogène. Les technologies évoluent aussi, en particulier l'électrolyse à haute température, avec des rendements deux à trois fois supérieurs aux autres technologies. Cela mérite, me semble-t-il, un soutien fort à la recherche pour accélérer les brevets et les innovations dans ce domaine. Ensuite, le stockage, point faible de l'électricité, est évidemment un axe important du développement de l'hydrogène. Les batteries issues de l'industrie automobile seront bientôt associées en série et nous disposerons également de produisant des batteries XXL, capables de stocker les surplus de production avant leur transformation par électrolyse.

En revanche, et c'est très surprenant, le couplage au nucléaire est à ce jour absent des intentions gouvernementales. On ne trouve aucun mot à ce sujet dans les différents plans hydrogène, certes certes élaborés avant la conversion au nucléaire du président Macron, révélatrice d'un sacrifice industriel et commercial pour de basses oeuvres politiciennes. Il est temps

économie circulaire mériterait davantage d'attention et d'intentions, pour contribuer, au passage, au verdissement de la filière gaz. D'autre part, les futurs réseaux de distribution doivent être construits en cohérence avec des schémas nationaux robustes et des emprises foncières

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cet hémicycle pour examiner la proposition de loi visant à assurer la qualité et la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, dont j'ai été à l'initiative, avec plus d'une centaine de mes collègues- 139 pour être exact -, de différents horizons politiques.

Cette pratique, dérogatoire au mode principal de déploiement de la fibre, par lequel l'opérateur d'infrastructures assure le déploiement dans son intégralité, présente deux singularités.

Le régulateur avait pourtant prévu un garde-fou en précisant que le recours automatique au mode Stoc ne serait valable qu'à la condition que les opérateurs commerciaux respectent strictement les règles de l'art.

Le mode Stoc a été un élément clé du déploiement massif et rapide de la fibre sur notre territoire. Alors que nous figurions parmi les plus mauvais élèves de l'Union européenne avant 2013, plus de 18 millions de Français sont désormais raccordés à cette technologie. Toutefois, ce succès ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. La situation actuelle n'est pas acceptable au regard des sommes engagées par l'État et les collectivités territoriales pour le déploiement de la fibre depuis 2013 dans le cadre du plan France Très Haut Débit

Le Gouvernement, l'Arcep et les opérateurs ont pris conscience du problème : dès 2019, un groupe de travail a été mis en place entre les opérateurs

un volet sous-traitance prévoyant une meilleure information de l'OC envers l'OI sur le recours à la sous-traitance et une limitation à deux du nombre de rangs de sous-traitants ; un

commerciaux de faire appel à des intervenants formés ; enfin, un volet sécurité, selon lequel l'OI doit s'assurer que chaque intervenant dispose des agréments nécessaires. Alors que ces nouveaux contrats auraient dû être mis en oeuvre avant la fin de 2020, ils n'étaient toujours pas appliqués sur une grande partie du territoire 2022. Face à cette inertie et à l'exaspération légitime des usagers et des élus locaux, j'ai déposé en juillet 2022 la proposition de loi qui vous est soumise Monsieur le ministre, dès votre nomination, en juillet dernier, vous avez exprimé votre volonté de vous saisir de ce sujet ; je salue votre engagement. Les opérateurs ont d'ailleurs promis de nouvelles mesures en septembre 2022.

Néanmoins, nous avons le droit de nous interroger sur la crédibilité de ces annonces comme sur la capacité de la filière à mettre rapidement en place les mesures promises depuis trois ans. trois ans. La fermeture du réseau cuivre étant désormais engagée, nous ne pouvons plus nous permettre de repousser les échéances. C'est la raison pour laquelle ce texte a été inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée.

L'article 1 de la proposition de loi vise principalement à clarifier la répartition des responsabilités entre opérateurs et à rappeler le rôle de garant de la qualité des raccordements souligne que le recours au mode Stoc relève d'un choix de l'OI pour rétablir un véritable principe de sous-traitance et met en place des outils pour assurer la bonne réalisation des travaux et la réparation des malfaçons. D'une part, il crée un guichet unique auprès de l'OI, chargé de traiter les difficultés de raccordement rencontrées par les usagers. D'autre part, il prévoit la remise systématique à l'utilisateur final, par l'intervenant chargé du raccordement, d'un certificat attestant de la conformité des opérations aux règles de l'art. L'utilisateur pourra également se prévaloir face aux opérateurs des stipulations des contrats de sous-traitance, lesquels devront intégrer des garanties en matière de qualité de raccordement et de contrôle.

Dans ces secteurs, déjà entièrement raccordables à la fibre et dans lesquels la transition de l'ADSL vers cette technologie va s'accélérer, il m'a semblé indispensable que la qualité des raccordements fasse l'objet d'une attention particulière. Le deuxième axe concerne plus spécifiquement les leviers à disposition des collectivités pour contrôler la bonne réalisation des raccordements dans les réseaux d'initiative publique La qualité des raccordements revêt en effet une importance supplémentaire dans ces zones, car les réseaux y sont déployés grâce aux deniers publics. L'article 2 prévoit notamment la remise à la collectivité porteuse du RIP des certificats attestant de la qualité des raccordements afin que celle-ci puisse vérifier la bonne réalisation des travaux. En l'absence de remise de ces certificats, la collectivité ne sera pas tenue de rémunérer l'opérateur pour les travaux de raccordement. C'est normal ! Le troisième levier concerne les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep. L'article 4 octroie au régulateur des télécommunications des pouvoirs spécifiques pour garantir la qualité des raccordements à la fibre à plusieurs égards. Il confère ainsi une base législative au pouvoir de police spéciale des communications électroniques que détiennent conjointement l'Arcep, le ministre en charge du numérique et l'Agence nationale des fréquences (ANFR). Il prévoit également la publication trimestrielle par l'Arcep d'indicateurs portant sur le niveau de qualité de service des réseaux fibre transmis par les opérateurs.

Enfin, le dernier levier concerne la protection des droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée de l'accès à internet. L'article 5 vise ainsi à renforcer cette protection par la création de trois nouvelles pénalités à l'encontre du fournisseur d'accès à internet, selon la durée de la panne : suspension du paiement de l'abonnement d'abord ; versement d'une indemnité à l'abonné par l'opérateur ensuite ; enfin, résiliation sans frais de l'abonnement par l'usager.

objectif n'est en aucun cas de remettre en cause le modèle actuel, mais bien de guider et d'accompagner les démarches de qualité en cours afin de mieux les traduire sur le terrain. À cet égard, j'invite les opérateurs à lire le texte. dans un état d'esprit d'équilibre avec la rapporteure de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, Patricia Demas, que je tiens à remercier pour son écoute, son implication et les compléments utiles qu'elle a apportés au texte initial. La qualité des réseaux fibre est La qualité des réseaux fibre est un sujet d'intérêt national qui ne saurait dépendre exclusivement du bon vouloir des acteurs économiques. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous

Je tiens à remercier mon collègue Patrick Chaize d'avoir déposé ce texte, qui apporte des solutions pragmatiques pour remédier aux désordres occasionnés dans le raccordement d'utilisateurs finaux à la fibre, en raison du recours à une chaîne de sous-traitance, souvent mal maîtrisée, dans le cadre du mode Stoc.

expression désigne un mode de réalisation des raccordements à la fibre par lequel l'opérateur d'infrastructure, responsable du réseau, confie la dernière partie du raccordement aux opérateurs commerciaux, qui font généralement eux-mêmes appel à d'autres prestataires. Alors que cette pratique était l'exception avant 2015, ce mode opératoire est devenu la règle. Nous avons tous constaté dans nos territoires

À l'aube de la fermeture du réseau cuivre, le raccordement final à la fibre optique est sans conteste le talon d'Achille du plan France Très Haut Débit. Il est dès lors de notre responsabilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la réussite de ce projet ambitieux, alors même que nous entrons dans sa dernière ligne droite. Face aux problèmes liés à la qualité des raccordements à la fibre, trois options s'offrent à nous. La première, privilégiée par le Gouvernement jusqu'à maintenant, consiste à négocier avec les opérateurs une solution contractuelle non prescriptive. Si ce mode d'action apparaît comme le plus souple, force est de constater qu'il est pour le moment insuffisant et qu'il n'a pas produit les résultats escomptés. La révision des contrats Stoc, engagée en 2020 grâce aux contrats dits Stoc II puis Stoc III, a permis des progrès, qui restent toutefois Le constat est clair : trois ans après le début des négociations, les engagements pris par les opérateurs peinent encore à être mis en oeuvre. La négociation avec la filière est indispensable, mais elle gagnerait à être encadrée et accompagnée par le législateur si nous souhaitons accélérer la montée en qualité des réseaux fibre et venir à bout des réticences de certains opérateurs. La deuxième option, la plus radicale, consisterait à mettre fin au mode Stoc et à charger l'opérateur d'infrastructure de la réalisation du raccordement, passant donc en mode OI. À première vue, il peut s'agir de la solution la plus évidente et je comprends que nombre d'acteurs, certains élus locaux notamment, aient pu l'avoir à l'esprit. Elle cependant à changer de plan au milieu de la bataille, alors que, depuis 2018, 20 000 locaux en moyenne sont raccordés chaque jour à la fibre. Changer de mode opératoire à ce stade risquerait de mettre un coup d'arrêt à ce déploiement, ce qui ne serait pas conforme à nos objectifs. La troisième option, à laquelle je souscris pleinement, consiste à mieux encadrer le mode Stoc. Cette solution pragmatique permet de répondre aux préoccupations des usagers et des collectivités sans pour autant renverser la table ni déstabiliser les dynamiques à l'oeuvre. à l'oeuvre. Le présent texte s'inscrit pleinement dans cette troisième voie d'équilibre. Je remercie Patrick Chaize et la commission de m'avoir accordé leur confiance Dans des délais restreints, j'ai entendu toutes les parties prenantes- opérateurs, régulateur, administrations centrales, élus locaux et usagers -et proposé à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable de reprendre plusieurs de leurs suggestions. J'en viens à présent

Conformément aux objectifs de Patrick Chaize, nous avons prévu, à l'article 1, que l'opérateur d'infrastructure confie la réalisation du raccordement à la fibre à l'opérateur commercial selon un mécanisme de priorité et sous réserve du strict respect des règles de l'art. Cette proposition pragmatique permet de conserver la volonté de l'auteur de garantir un principe de sous-traitance, en rappelant que la mise en oeuvre du mode Stoc relève d'un choix de l'opérateur d'infrastructure, tout en préservant l'équilibre des contrats de sous-traitance en cours. Avec le même objectif, la commission a souhaité renforcer le caractère opérationnel du guichet unique pour prendre en charge les difficultés de raccordement à la fibre rencontrées par les utilisateurs.

Ce guichet unique a suscité des réactions différentes chez les usagers, les opérateurs et le Gouvernement. Si tout le monde s'accorde sur son utilité, la définition de ses modalités opérationnelles fait débat.

Enfin, la commission a modifié l'article 3, qui interdit le recours au mode Stoc dans certaines zones du territoire, pour en affiner le périmètre d'application afin de prendre en compte la fermeture du réseau cuivre et restreindre l'interdiction aux raccordements longs et complexes, manière à limiter les atteintes à la liberté d'entreprendre. Le deuxième axe des travaux de la commission a été de consolider les exigences de qualité et de contrôle applicables aux raccordements. Nous avons prévu, à l'article 1, l'élaboration d'un socle d'exigences minimales de qualité, que les contrats et les cahiers des charges liant les opérateurs commerciaux et leurs sous-traitants devront respecter. Nous avons également introduit une obligation de labellisation de tout intervenant chargé de réaliser un raccordement à la fibre, selon un référentiel national. nous avons consacré dans la loi la réalisation systématique d'un compte rendu d'intervention pour permettre à l'opérateur d'infrastructure et à l'utilisateur de vérifier la bonne réalisation du raccordement.

à renforcer les moyens de contrôle des élus locaux, souvent démunis face aux malfaçons dans le raccordement final. Le troisième et dernier axe des travaux de la commission a été d'assurer le caractère opérant des dispositifs.

À l'article 5, qui ouvre de nouveaux droits aux consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet, nous avons, d'une part, amélioré l'articulation dans le temps des sanctions

tous ces ajustements de bon sens, qui résultent d'un travail approfondi de concertation avec tous les acteurs, s'inscrivent pleinement dans l'esprit du texte présenté par Patrick Chaize tout en consolidant sa portée et son caractère opérationnel. Vous l'aurez compris, face aux dysfonctionnements dans le raccordement des utilisateurs finaux à la fibre optique, il n'existe pas de solution miracle donnant satisfaction à l'ensemble des intervenants. Il y a pourtant urgence à agir pour assurer la pérennité et la qualité des raccordements. Le texte de la commission est une proposition ambitieuse et équilibrée, mais nous avons conscience qu'elle est aussi perfectible.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à remercier Patrick Chaize pour le dépôt de cette

par le secteur privé, 25 % par les collectivités territoriales et 10 % par l'État. C'est également l'un des chantiers

Dans leur minorité, les problèmes sont liés aux opérateurs commerciaux. C'est là le sujet de la proposition de loi que nous allons discuter. En raison

ou de coupures sauvages : les sous-traitants des opérateurs commerciaux se présentent devant une armoire pour opérer le raccordement d'un client dans des temps très contraints et le font parfois de manière non appropriée ou au détriment d'usagers déjà raccordés.

à ce que l'opérateur commercial installe le dernier kilomètre, en lien avec son client, sauf s'il le fait dans des conditions de qualité dégradées.

(Amii), les opérateurs ont pris des engagements pour permettre ce développement. Dans les autres, les collectivités locales se sont emparées du sujet à bras-le-corps afin d'apporter les mêmes services dans les territoires ruraux. Sur le papier, la répartition était équilibrée et a bien fonctionné, comme on peut le constater dans un territoire que je connais bien, l'Aisne, qui est l'un des départements ruraux les mieux fibrés de France. Cependant, certains élus locaux ont fait remonter à plusieurs reprises des difficultés de raccordement. Ici, une personne est mécontente de constater que son voisin est bien raccordé tandis

À l'heure du tout-numérique, cette situation, lorsqu'elle perdure, peut être très pénalisante tous secteurs confondus. Aussi, au regard de cette situation, nous saluons le travail de notre collègue Patrick Chaize, auteur de cette proposition de loi, ainsi que celui de la rapporteure. Ce texte prévoit des mesures concrètes pour encadrer la sous-traitance et protéger les usagers. Généralement, le problème, c'est le raccordement de la fibre jusqu'au domicile de l'abonné, dans la mesure où ce raccordement s'effectue dans une armoire dite spaghettis.

Le mode Stoc, régulièrement utilisé par les opérateurs d'infrastructure, implique l'intervention de sous-traitants, de sorte que l'on s'éloigne de la chaîne initiale ayant déployé le réseau. Il est donc nécessaire de poser clairement le principe de responsabilité des opérateurs d'infrastructure tout en apportant des garanties aux abonnés. Cela passe par la mise en place d'un socle d'exigences minimales, lequel est donc bienvenu dans ce texte. Les techniciens qui interviennent doivent en effet disposer d'une formation adéquate pour effectuer « dans les règles de l'art » la réparation ou le raccordement requis.

Le compte rendu d'intervention est la première étape pour garantir ce suivi. Il faudra également veiller à ce que les contrôles soient effectifs et suivis d'effet. Nous espérons ainsi que l'Arcep disposera des moyens financiers suffisants pour mener à bien cette mission.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fibre optique est devenue le principal réseau d'accès à internet pour les Français : le taux de locaux raccordables approche aujourd'hui les Mais si le déploiement de la fibre progresse bien à l'échelle nationale- cela a été dit -, de fortes disparités régionales demeurent. Selon le rapport de France Stratégie de 2023, certains départements à dominante rurale dépendent toujours à plus de 25 % du réseau cuivre. Je le souligne ici, et je sais que nous partageons cette analyse, le non-accès à la fibre porte gravement atteinte à un aménagement équilibré du territoire et constitue une rupture d'égalité qui ne peut être tolérée. Le cap de 2025 a été fixé pour la généralisation de la fibre afin de garantir son accès à tous les usagers. Il est de notre responsabilité, ici, au Sénat, de nous assurer du respect de cet objectif. Nous avons tous en

dès 2019 en vue d'améliorer l'exploitation des réseaux et de résoudre les difficultés. Manifestement, les démarches entreprises par les opérateurs en concertation avec le Gouvernement sont insuffisantes, comme l'a souligné l'auteur de ce texte, Patrick Chaize, que

Elle doit permettre d'améliorer le déploiement du plan France Très Haut Débit et de limiter les difficultés et les dysfonctionnements liés à ces raccordements. Ce texte apportera des outils législatifs pour réguler et contrôler les opérateurs et leurs sous-traitants, pour renforcer les pouvoirs de l'Arcep et mieux protéger les consommateurs, et ainsi rassurer les collectivités

à la fibre tout en veillant à ne pas ralentir le déploiement de cette technologie, à deux ans de l'achèvement du plan et alors que la fermeture du réseau cuivre est imminente. Pour le groupe Écologiste- Solidarité et Territoires, il est essentiel de renforcer la garantie de la qualité du raccordement

Par ailleurs, les collectivités, en particulier dans les zones rurales, ont été affectées par la mauvaise gestion du déploiement de la fibre, car c'est vers elles que se sont souvent tournés ceux qui ont rencontré des difficultés de connexion. Il est donc essentiel de consulter davantage les élus locaux et, après un constat de carence dans les zones d'initiative privée, de prévoir de nouveaux appels à manifestation d'intérêt. Pour la protection des consommateurs, notre groupe proposera un amendement travaillé avec l'UFC-Que Choisir visant à Choisir visant à modifier les seuils de sanction en cas d'interruption du service d'accès à internet. Une protection efficace des consommateurs paraît nécessaire, car la perte d'une connexion à internet a des conséquences

Les objectifs fixés étaient les suivants : le raccordement de 100 % des 35 millions de logements et locaux à usage professionnel, dont 80 % en fibre optique jusqu'à l'abonné en 2022, et la généralisation de la fibre optique en 2025. en sorte que, d'ici à deux ans, tous les Français, notamment ceux qui habitent en zone rurale, puissent bénéficier d'une connectivité numérique performante, chez eux comme sur leur lieu de travail. Pour rappel, il y a dix ans, le plan prévoyait initialement 20 milliards d'euros d'investissements publics et privés, dont 3,3 milliards de subventions de l'État à destination des collectivités locales dans les zones dites non conventionnées. Dans un rapport publié en janvier 2017, la Cour des comptes avait toutefois substantiellement réévalué le coût du plan à 35 milliards d'euros, et estimé que si l'objectif intermédiaire d'une couverture de 50 % du territoire était atteint, l'objectif en matière de très haut débit fixé pour 2022 semblait compromis par l'insuffisance du co-investissement privé. Dans le cadre du plan de relance présenté en septembre 2020, le Gouvernement a amplifié son effort et mobilisé 420 millions d'euros pour soutenir les collectivités locales qui en avaient le plus besoin, n'ayant pu encore viser la généralisation de la fibre. Je pense à la Bretagne, à Mayotte et à l'Auvergne à titre d'exemples. Quel constat faisons-nous aujourd'hui ? L'objectif d'une couverture de 80 % du territoire en fibre optique était quasi atteint au 31 décembre 2022, ce qui place la France à la tête des pays les plus fibrés en Europe.

à l'horizon 2026. S'il est incontestable que la France a mis en oeuvre une dynamique puissante de déploiement de la fibre, force est aussi de constater- c'est l'objet de cette proposition de loi -que des difficultés opérationnelles sont apparues, parfois de manière intolérable, notamment pour les collectivités territoriales qui s'en sont fait l'écho. En effet, le modèle de déploiement de la fibre repose principalement sur la sous-traitance- ce qu'on appelle le mode Stoc -, laquelle subit une forte pression sur les prix de la part des donneurs d'ordre. Or la sous-traitance ne permet pas un contrôle optimal de la formation des techniciens chargés d'effectuer les raccordements, ce qui entraîne des malfaçons non seulement sur le réseau, mais aussi parfois sur les infrastructures situées à proximité, à l'instar des tableaux électriques ou des réseaux de gaz. Si l'Arcep recommande un plafond de deux rangs de sous-traitance, l'Autorité indique avoir observé des opérations portant à cinq, voire à six, le nombre de rangs de sous-traitance. Les points de mutualisation situés en pleine rue concentrent les branchements des câbles de fibre optique et les difficultés opérationnelles

à la description alarmante de la situation en matière de raccordement des abonnés à la fibre optique effectuée dans l'exposé des motifs de la proposition de loi de juillet 2022, les acteurs de la filière ont pris pleinement conscience des difficultés rencontrées par certains usagers, de leur insatisfaction et des légitimes préoccupations des élus locaux, de même que de la vigilance des parlementaires sur ce sujet. Face au tableau parfois sombre qui est fait du déploiement de la fibre, les opérateurs se devaient de réagir. En septembre dernier, un plan d'action a donc été décidé par les acteurs de la filière, qui repose notamment sur la prise de photos avant et après l'opération, lesquelles sont jointes au compte rendu d'intervention, et sur la remise en état des points de mutualisation. La Fédération française des télécoms vient aussi de publier des grilles de compétences à destination des donneurs d'ordre, qu'il s'agisse des opérateurs commerciaux ou des opérateurs d'infrastructure, et de leurs prestataires. Le référentiel concernant les sous-traitants porte notamment sur la formation de leurs techniciens, sur les règles de sécurité et d'ingénierie pour les travaux optiques ou sur les bonnes pratiques lors de travaux chez le client.

Celle-ci a d'ores et déjà produit des effets, manifestement dans le bon sens, puisque le Gouvernement a obtenu un certain nombre d'engagements et de concessions de la part des opérateurs. Il nous appartient donc de donner des signes de notre volonté d'agir. À cet égard, et même si certains peuvent juger raisonnable de laisser du temps à la filière pour poursuivre la résolution des dysfonctionnements constatés en juillet 2022, ce texte est

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le numérique, qu'on appelait il y a encore une décennie les nouvelles technologies de l'information et de la communication, connaît un essor considérable et conditionne désormais notre développement économique et notre vie sociale. Le numérique prend appui sur le triptyque que constituent les infrastructures, les services et les usages. Le déploiement des infrastructures permettant le haut débit est un préalable et une nécessité pour permettre aux opérateurs et aux sociétés dédiés de proposer des services et aux utilisateurs de s'approprier des usages dont on n'imaginait pas l'étendue il y a encore quelques années. Ce déploiement vital des infrastructures s'effectue en un temps record si on le compare au déploiement d'autres infrastructures tout aussi déterminantes. Ainsi, sans parler du réseau ferroviaire, qui a quadrillé la France en quatre-vingts ans, le réseau électrique s'est déployé sur un bon demi-siècle, de même que le réseau d'adduction d'eau potable.

du plan France Très Haut Débit en 2013, sous François Hollande, s'inscrivait dans la continuité de la volonté d'un État stratège, qui visait à couvrir l'intégralité du territoire en très haut débit en moins d'une décennie. Ce plan, il faut le reconnaître, est un succès et le rythme des déploiements s'est accéléré. Ainsi, en 2022, ce sont 4,7 millions de foyers supplémentaires

Malheureusement, et c'est l'objet de cette proposition de loi, la qualité des raccordements finaux n'est pas toujours au rendez-vous, ce qui entache le succès du plan France Très Haut Débit et génère la colère et la frustration de bon nombre de nos concitoyens. Il semble en effet que nous ayons confondu vitesse et précipitation, et que l'atteinte d'objectifs chiffrés l'ait emporté sur la qualité du raccordement final proposé à l'usager. Les faits sont désormais objectivés et le mode de sous-traitance à l'opérateur commercial, censé éviter au domicile de l'usager la double intervention de celui qui livre l'infrastructure de raccordement final et de celui qui propose l'ouverture du service à un opérateur, a démontré ses limites. Les vents de l'ubérisation de la sous-traitance et du partage non équitable de la valeur ont également soufflé sur le secteur des télécommunications, comme sur bien d'autres, hélas Dès lors, face aux dysfonctionnements constatés, fallait-il légiférer ou se contenter de contester, d'interpeller les acteurs, dont les opérateurs, de faire les gros yeux et d'en appeler au régulateur ?

d'établir un parallèle avec un sujet qui nous a mobilisés il y a deux ans : la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Le Sénat- souvenez-vous-en -, dans le cadre d'une mission d'information, avait mis en évidence cet angle mort de nos politiques publiques,

L'objectif de nous voir toutes et tous connectés se heurte à celui de la rentabilité et à la politique du chiffre, qui provoque de nombreux désagréments sur le terrain. Malfaçons, raccordements ratés, débranchements intempestifs : les collectivités et les usagers font face à de lourdes difficultés lorsqu'il s'agit de désigner un responsable à ces manquements. Selon l'Avicca, qui regroupe les collectivités engagées dans le numérique, près de 75 % des raccordements réalisés en mode Stoc présentent des défauts. Le phénomène n'est pas nouveau et les appels à la vigilance des opérateurs sont récurrents, mais les contrats Stoc V1, V2 et V3 n'y ont rien changé. La proposition de loi que nous examinons a le mérite, dans un contexte où les usagers, les installateurs ou les installations font l'objet d'un mauvais traitement, de mieux encadrer le déploiement par les opérateurs privés jusqu'alors guidés par la rentabilité, la quantité des foyers raccordés primant la qualité du réseau. Je salue le travail de nos collègues Patrick Chaize et Patricia Demas,

La médiatrice des communications électroniques évoquait « les naufragés de la fibre » dans un rapport de 2021, en soulignant les dysfonctionnements occasionnés par des installations bâclées. Alors que le réseau cuivre, dit réseau historique d'Orange, devrait être démantelé d'ici à 2030, il est légitime d'exiger des opérateurs des garanties afin de permettre le basculement vers la fibre dans les meilleures conditions pour les usagers. La sous-traitance, qui devait être dérogatoire pour le raccordement final de la fibre au domicile, est devenue la règle, nous l'avons constaté. Or c'est précisément cette sous-traitance en cascade

à celles et à ceux qui subissent une forme d'ubérisation qui les pousse à réaliser toujours plus de raccordements, sans en avoir véritablement les moyens, et qui sont surtout mal rémunérés. La mise en place d'un guichet unique pour assurer la prise en charge des difficultés sur le terrain, d'un certificat de conformité sur le modèle des raccordements au gaz et d'un contrat de sous-traitance élaboré par l'opérateur d'infrastructure et soumis à l'Arcep participe des améliorations nécessaires et susceptibles de corriger la situation existante. Les droits des consommateurs sont par ailleurs renforcés- c'est important -et des sanctions sont prévues en cas d'interruption du service. Cette proposition de loi pourrait aller plus loin en remettant en cause le modèle même du déploiement de la fibre. Je pense notamment à ce que nous avons su faire pour nos réseaux de télécommunications historiques ou pour celui du gaz et de l'électricité- permettez-moi d'y penser ! ERDF, GRDF ou France Télécom : ces noms résonnent comme des vestiges après tant d'années de déstructuration et de privatisation Les opérateurs publics sont pourtant des gages de réussite, de durabilité et d'efficacité pour un déploiement qui est avant tout un enjeu d'intérêt général, À l'heure où nous donnons au numérique une place de plus en plus importante dans nos vies, où la dématérialisation poursuit son chemin, y compris en matière de services publics, cette proposition de loi, grâce aux objectifs qu'elle affiche, participe de la réduction de la fracture numérique, alors que l'on sait que 13 millions de nos que 13 millions de nos concitoyens sont en situation d'illectronisme. Parce que ce texte permettra une amélioration concrète, visible et attendue sur le terrain, le groupe CRCE le votera.

réalisés jusqu'à l'abonné tout en évitant la dégradation des équipements des réseaux optiques. En effet, de nombreux dysfonctionnements sont observés au quotidien par les administrés, qu'il s'agisse de coupures répétées ou de la fragilisation du réseau. Ces problèmes sont liés au recours à la sous-traitance dite Stoc, c'est-à-dire à la sous-traitance à l'opérateur commercial du raccordement des abonnés à la fibre.

Mais force est de constater que de nombreux problèmes sont relevés depuis l'accélération du déploiement de la fibre sur notre territoire. C'est un sujet dont je discute souvent avec mes collègues du groupe Union Centriste, notamment avec Évelyne Perrot, que j'associe à mes propos. Cette technologie doit pourtant répondre à un besoin grandissant de communication et de numérisation du quotidien des Français. Je pense particulièrement à l'accès aux démarches administratives, qui sont désormais quasiment toutes dématérialisées, que ce soit en matière d'état civil, de sécurité sociale, de scolarité, d'impôts ou encore d'accès au logement.

Un accès stable à internet est désormais une nécessité et la fibre optique présente bien des avantages grâce à sa grande capacité de transport d'informations, à ses interférences réduites et à sa meilleure durée de vie. À ce jour, c'est la technologie qui permet d'atteindre les meilleurs débits internet. La France avait très bien commencé son pari numérique, puisque 34 millions de foyers, d'entreprises et d'administrations ont été rendus raccordables à la fibre optique en 2022. Mais pour que la fibre soit une réalité pour tous, de très importants travaux ont été et sont encore nécessaires.

la mairie devient naturellement le bureau des pleurs, le réceptacle des reproches et l'endroit privilégié où des consommateurs excédés espèrent trouver une réponse à leurs difficultés. Les différentes initiatives des opérateurs pour répondre aux attentes des élus et des administrés, qu'il s'agisse de la création du mode Stoc V2 en 2020 ou du plan qualité en 2022, n'ont pas permis de rétablir complètement la situation. Après une longue période de patience, cette situation n'est plus supportable : de nouveaux engagements doivent être pris par les différentes parties, et ce d'autant plus que l'objectif du Gouvernement est de généraliser la fibre optique sur l'ensemble du territoire d'ici à 2025.

Le texte prévoit que les contrats de sous-traitance devront être conformes à un modèle élaboré par l'opérateur d'infrastructure, soumis à l'avis préalable de l'Arcep et opposable par les usagers. Chaque intervenant chargé d'effectuer un raccordement à la fibre remettra à l'abonné un certificat attestant de la conformité des travaux réalisés au cahier des charges. Ces mesures viennent utilement clarifier le mode de sous-traitance choisi et contribuent à garantir la transparence nécessaire au bon déroulement des travaux de raccordement. texte vise également à renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep, ainsi que les droits des consommateurs en cas d'interruption prolongée du service d'accès à internet. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat a, suivant en cela les orientations de sa rapporteure- que je salue

Il suffit d'en parler autour de nous pour constater le ras-le-bol général : la fibre est devenue un sujet de crispation du quotidien. Alors qu'internet est aujourd'hui un outil indispensable, y compris pour accéder aux services publics les plus essentiels, les coupures à répétition, les erreurs de raccordement et les malfaçons du réseau fibré sont particulièrement mal vécues.

La proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize, que nous sommes plusieurs à avoir cosignée au sein du groupe du RDSE, prévoit des solutions pour pallier les dysfonctionnements qui surviennent dans le raccordement final de l'usager. Cette responsabilité a été sous-traitée par l'Arcep aux opérateurs commerciaux et aux fournisseurs d'accès à internet. Les contrats de sous-traitance dits Stoc sont une exception, une dérogation devenue la règle. Ils ont sans aucun doute permis le déploiement rapide de la fibre et son succès commercial,

Sans remettre en cause l'équilibre actuel et la dynamique du déploiement de la fibre, le texte issu des travaux de la commission comporte des pistes d'amélioration auxquelles nous souscrivons. Tout d'abord, la proposition de loi précise que, si le raccordement est confié en priorité à l'opérateur commercial, c'est à condition qu'il respecte strictement les règles de l'art. Tout en rappelant que l'opérateur d'infrastructure est responsable de son réseau, nous garantissons ainsi la stabilité des contrats de sous-traitance en cours. Ensuite, tout en restant la norme, la sous-traitance aux opérateurs commerciaux serait interdite pour les raccordements longs et complexes dans les zones déjà fibrées, dans les communes où la fermeture du réseau cuivré est engagée et en cas de simple changement de fournisseur d'accès à internet par un abonné déjà raccordé. Ces précisions devraient permettre de concentrer le mode Stoc sur le déploiement massif et rapide de la fibre, tout en garantissant un niveau de qualité optimal dans les zones les plus tendues et dans les cas les plus complexes.

et le Gouvernement, sont opposés à ce texte, notamment à certains de ses aspects : ils considèrent que cette proposition de loi pourrait conduire à la déstabilisation d'un modèle qui a fait ses preuves. Confier le raccordement final à l'opérateur d'infrastructure entraînerait en effet une réorganisation de la filière et, peut-être, un ralentissement du déploiement de la fibre.

liés à un recours parfois mal maîtrisé à la sous-traitance dans le cadre du mode de sous-traitance aux opérateurs commerciaux, dit mode Stoc. Le déploiement de la fibre optique en France est un enjeu majeur pour l'aménagement du territoire, le développement économique et social du pays, ainsi que pour la compétitivité de nos entreprises. C'est également un enjeu de développement durable, puisque la fibre optique est une technologie plus économe en énergie que les technologies existantes et qu'elle favorise la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre.

D'un point de vue européen, le déploiement de la fibre optique en France se fait à un très bon rythme, puisque la part de la fibre a doublé en deux ans, passant d'environ 24 % en 2019 à 46 % en 2021.

De cette couverture globale et qualitative dépendra la réussite finale du plan France Très Haut Débit. Dès lors, la présente proposition de loi, examinée et amendée par notre Haute Assemblée, sous la férule de notre rapporteure Patricia Demas, permet de fixer un cadre de mise en oeuvre du mode Stoc, de clarifier la répartition des responsabilités, de renforcer les contrôles de la qualité des raccordements et de protéger les droits des usagers en cas d'interruption des services internet. Dans le détail, il s'agit notamment de rappeler la responsabilité de l'opérateur d'infrastructure dans le choix du mode de réalisation des raccordements et son rôle de garant de la qualité des travaux et d'instaurer un guichet unique assurant la prise en charge des difficultés de raccordement. Il s'agit également d'interdire le mode Stoc dans les zones fibrées et dans les communes dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre est engagée. Il s'agit aussi d'accroître les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'Arcep sur tous les opérateurs intervenant sur le réseau. Il s'agit enfin de renforcer les droits des consommateurs face aux effets des coupures prolongées d'accès à internet et aux débranchements sauvages, tout en protégeant les opérateurs commerciaux contre d'éventuels abus des consommateurs.

Comme toujours, ceux qui sont en première ligne face aux difficultés des administrés- les maires -se sont largement mobilisés, en particulier en interpellant directement l'Arcep. C'est pourquoi la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize va dans la bonne direction. en particulier à l'article 5 relatif au renforcement des droits des consommateurs en cas d'interruption d'un service d'accès à internet, qui permettra de mieux protéger les Français, notamment les plus vulnérables, trop souvent démunis

d'un lieu commun, il convient de rappeler que le numérique, et internet en particulier, s'est introduit au coeur de la vie des Français depuis une vingtaine d'années. seulement le télétravail, la consommation de biens et de services sur des sites marchands, mais également le maintien du lien avec nos proches, le développement et le partage de nos passions, l'accès à l'information, l'apprentissage ou encore l'accès aux droits sur les plateformes de l'administration publique. Le numérique permet l'émancipation des individus, mais cet effet émancipateur est à double tranchant plus la digitalisation de la société avance, plus ceux qui restent sur le bord de la route du numérique se retrouvent progressivement en situation d'exclusion. Ainsi, notre vigilance doit être toute particulière s'agissant de la fracture numérique, aussi bien celle du premier degré, qui concerne l'accès matériel, physique au numérique, que celle du second degré, qui concerne les usages, ceux des 16 millions de personnes en situation d'illectronisme, un nombre qui ne cesse d'augmenter. d'augmenter. L'éloignement du numérique concerne davantage nos concitoyens les plus précaires, les moins diplômés, ceux pour qui l'accès à l'information et le recours à leurs droits sont un impératif, notamment à l'heure de l'administration 100 % dématérialisée.

Or nous le constatons aujourd'hui en tant qu'élus locaux, mais également en tant que consommateurs : la dégradation de la situation est telle qu'elle nécessite, outre une prise de conscience, un engagement fort, dût-il passer par la loi.

Cette situation, qui perdure malgré la signature en 2021 du contrat Stoc V 2, lequel est destiné à mieux encadrer les pratiques et à régler les nombreux dysfonctionnements, est aujourd'hui inacceptable.

Le choix de ce mode de gestion, que nous n'allons pas remettre en cause aujourd'hui, ne saurait cependant en aucune manière justifier une quelconque dégradation de la qualité du réseau. Alors que, à terme, la fibre optique jusqu'à l'abonné sera l'unique moyen d'accès aux services numériques en très haut débit, l'exigence de qualité, en termes de raccordement ou d'exploitation, appelle un véritable effort de long terme pour que soit assurée une maintenance des infrastructures. À cet égard, nous sommes aujourd'hui le relais de l'exaspération de nos territoires, qui multiplient les motions contre le plan d'extinction du cuivre prévu tant que les difficultés de raccordement à la fibre ne seront pas résorbées et qui plaident pour un entretien sérieux des infrastructures en place, lesquelles se dégradent dangereusement. Dans la Sarthe, département dont je suis élu, ces motions datent de la semaine dernière ! Aussi, et sans renier les efforts d'ores et déjà fournis par l'Arcep en synergie avec les opérateurs à travers son plan qualité, la

à la charge du responsable du réseau, ce qui permettra d'assurer un service après-vente rapide. Elle instaure des obligations pour l'intervenant, qui devra fournir un compte rendu d'intervention, ainsi qu'un certificat de conformité au cahier des charges qui lui est imposé. Elle fait par ailleurs en sorte que l'Arcep puisse jouer efficacement son rôle. Enfin, elle sécurise les droits du consommateur final, qui ne doit pas pâtir de la situation actuelle et rester démuni lorsqu'il est privé de services, alors même qu'il paie un abonnement.

proposition de loi.

La France s'est fixé des objectifs ambitieux pour développer la fibre optique dans le cadre du plan France Très Haut Débit. D'ici à 2026, l'intégralité de la population et des entreprises devra être raccordée. Alors que que près de 80 % de la population est d'ores et déjà raccordée, nous sommes assurément l'un des pays d'Europe les plus performants en matière de déploiement même si, ces derniers temps, une ombre au tableau atténue cette réussite : les raccordements FttH ( - fibre jusqu'à l'abonné) effectués sur les derniers mètres par les opérateurs commerciaux et leurs sous-traitants sont devenus une véritable jungle du fait de la souplesse du mode Stoc. Détérioration des équipements, brassages inextricables, non-respect des routes optiques, locaux abîmés et laissés ouverts, dépôts sauvages de matériel dans les, abonnés débranchés au profit d'autres usagers : la liste des malfaçons ne cesse de s'allonger.

Cette situation est inadmissible au regard des montants colossaux engagés pour déployer la fibre et entraîne un véritable gâchis d'argent public. Monsieur le ministre, je vous ai interpellé le mois dernier à ce sujet. Vous m'aviez alors répondu que le problème était probablement dû à l'accidentologie du réseau en lui-même. Or les dégradations existent partout, y compris sur des réseaux considérés comme peu accidentogènes. Il est évident qu'elles résultent des mauvaises pratiques des opérateurs commerciaux et de leurs sous-traitants permises par le mode Stoc. Cette exception à la française, qui devait initialement être dérogatoire, mais qui est devenue la norme, a clairement montré ses limites. limites. Les opérateurs ont certes pris des engagements pour que cessent ces détériorations. Des formations labellisées ont également été mises en place et un plan de reprise des points de mutualisation dégradés a été lancé, mais force est de constater qu'aucune amélioration ne se fait ressentir. La présidente de l'Arcep a elle-même reconnu publiquement qu'il n'y avait aucune véritable avancée malgré les mesures mises en oeuvre. Il faut donc regarder la réalité en face et conclure à l'échec du mode Stoc dans sa version actuelle. L'adoption de mesures coercitives est nécessaire pour corriger le tir, la méthode contractuelle n'ayant pas suffisamment porté ses fruits depuis sa mise en oeuvre en 2018. Il est donc temps de mettre les opérateurs commerciaux face à leurs responsabilités. Tel est précisément l'objet de la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize, que je ne peux que remercier pour son initiative. J'y souscris en tout point et je partage le constat établi : ce n'est qu'en encadrant le recours à la sous-traitance, en clarifiant la responsabilité de chacune des parties prenantes, en renforçant les contrôles

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à clarifier les modalités de réalisation des raccordements à la fibre et les obligations respectives des opérateurs il tend à préciser que les exigences de qualité et les obligations de labellisation des intervenants, de réalisation d'un compte rendu d'intervention et de remise d'un certificat de conformité s'appliquent aux travaux de raccordement, peu importe le mode opératoire retenu. Cette précision a pour objet de garantir l'application de ces dispositions aux cas où l'opérateur d'infrastructure effectue lui-même des opérations de raccordement. Ensuite, il vise à compléter utilement le dispositif en instituant un certificat qui sera remis à l'utilisateur final en cas d'échec de raccordement. objet de clarifier l'articulation entre les dispositions de l'article 1, qui prévoient l'opposabilité du contrat de sous-traitance par l'utilisateur final, et les sanctions qui peuvent être prononcées en cas d'interruption du service d'accès à internet en application de l'article 5.

Cet amendement vise à obliger l'opérateur commercial, lorsqu'il annule une commande de raccordement, à communiquer à l'opérateur d'infrastructure la raison à l'origine de ce revirement. Actuellement, dans un tel cas de figure, l'opérateur commercial ne documente pas systématiquement la raison de l'annulation auprès de l'opérateur d'infrastructure, ce qui empêche ce dernier de résoudre un problème relevant potentiellement de sa responsabilité.

un réseau numérique installé, avec un boîtier sur lequel la fibre optique peut être raccordée. Dans les faits, les raccordeurs de fibre optique n'interviennent pas forcément sur ce boîtier, parce qu'ils n'ont aucune obligation de le faire.

élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau ». Il s'agit par exemple des pylônes, des gaines, des chambres de tirage, des regards,

Depuis 2016, le gestionnaire d'infrastructures d'accueil doit faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, comme le réseau de fibre optique. Cet accès doit être fourni selon des modalités et dans des conditions équitables et raisonnables, et fait généralement l'objet d'une convention passée entre l'opérateur de communications électroniques et le gestionnaire de l'infrastructure d'accueil. Les infrastructures d'accueil peuvent être nécessaires à la réalisation du raccordement à la fibre d'un utilisateur final. Or il arrive qu'elles fassent l'objet de malfaçons ou de dégradations de la part des intervenants chargés d'effectuer un raccordement à la fibre. Par cet amendement, il s'agit donc de préciser que les exigences tendant à assurer la qualité de la réalisation des raccordements à la fibre s'appliquent également à l'utilisation des infrastructures d'accueil nécessaires à cette opération.

adopté, l'amendement n° 7 rectifié compléterait judicieusement le dispositif en garantissant mieux la qualité des raccordements en partie privative dans les logements récents, qui sont déjà équipés d'un réseau numérique.

la position du Gouvernement sur cet article 1 est assez prévisible et lisible. Il vise cette fois-ci les alinéas 4 et 5, qui concernent le guichet unique, et tend à préserver la relation entre l'usager, l'utilisateur et l'opérateur commercial.

Avis défavorable. Il y a un hiatus entre le dispositif de l'amendement, qui vise à supprimer l'obligation de labellisation des intervenants chargés d'effectuer le raccordement introduite en commission, et l'objet, qui indique que la modification n'est que rédactionnelle. La labellisation des intervenants est un prérequis nécessaire à la montée en qualité de la filière et de la sous-traitance.

Cet amendement vise à étendre ces obligations à l'hypothèse où ce dernier est amené à intervenir de nouveau pour réparer un raccordement défectueux, c'est-à-dire dans le cadre d'une opération dite de service après-vente. L'objectif est de permettre à l'opérateur d'être informé de toute intervention, quelle qu'elle soit, et du bilan de cette intervention, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. L'idée selon laquelle l'opérateur d'infrastructure doit avoir connaissance de ce qui se passe sur le réseau afin d'être en mesure de régler dans les meilleurs délais d'éventuelles défaillances me semble être un principe de bon sens. J'ajoute que, lorsque les raccordements à la fibre optique seront terminés sur l'ensemble du territoire, l'intervenant réalisera principalement des opérations de service après-vente. Il convient donc d'anticiper dès à présent cette future étape.

est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à clarifier le champ d'application des dispositions prévoyant la réalisation d'un compte rendu d'intervention et la remise d'un certificat de conformité pour les opérations de raccordement. à préciser que ces obligations s'appliquent également lorsqu'une nouvelle intervention est nécessaire, par exemple après un échec de raccordement.

et tend à créer un registre des interventions de raccordement d'utilisateurs finals au réseau à très haut débit en fibre optique. Celui-ci permettra de responsabiliser les opérateurs commerciaux, ainsi que leurs sous-traitants, et favorisera une meilleure traçabilité des interventions au bénéfice des opérateurs d'infrastructure et des autorités compétentes.

Il est prévu que celui-ci soit accessible, d'une part, à l'opérateur d'infrastructure, et ce afin de faciliter le contrôle des interventions de raccordement survenant sur son réseau, et, d'autre part, aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux autorités détentrices aux autorités détentrices du pouvoir de police des communications électroniques. S'il était adopté, cet amendement compléterait utilement l'article 1 et permettrait de mieux asseoir les dispositions de l'article 4, qui renforcent les pouvoirs de contrôle de l'Arcep en matière de qualité des raccordements.

premier alinéa prévoit que l'opérateur devra indiquer, à la fois pour les logements individuels et les logements collectifs, le point de raccordement le plus viable économiquement pour le propriétaire du bâtiment. Le deuxième alinéa indique que les travaux de raccordement et de mise en éligibilité commerciale doivent être achevés dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition par le propriétaire de l'adduction au réseau physique très haut débit. Enfin, le troisième alinéa concerne les potentiels travaux de raccordement d'adduction nécessaires aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, qui doivent être proposés et gérés par l'opérateur d'infrastructure. Ces trois précisions nous semblent nécessaires. Quel est l'avis de la commission ? Cet

Depuis la fin du service universel, Orange n'a plus l'obligation de raccorder au cuivre les logements neufs. Des usagers se retrouvent donc parfois sans solution d'accès au réseau en attendant d'être raccordés à la fibre. Je suis attentive au problème soulevé et je partage l'objectif d'assurer le raccordement à la fibre de ces locaux dans des délais raisonnables. Cependant, il me semble que, tel qu'il est rédigé, cet amendement est susceptible d'avoir d'importantes incidences incidences financières pour les opérateurs d'infrastructure et de désorganiser les déploiements en cours. Faute de pouvoir précisément en évaluer les conséquences et le caractère opérationnel, je m'en remets à l'avis du Gouvernement. Quel est l'avis du Gouvernement

Ce texte prévoit des mesures concrètes pour assurer la pérennité du réseau à très haut débit en fibre optique, qui est vital pour les citoyens et les acteurs socio-économiques, en particulier dans les zones rurales, où l'accès au réseau numérique a vocation à compenser l'éloignement des services publics. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, que j'ai l'honneur de présider, a adopté ce texte à l'unanimité, le 12 avril dernier, tout en l'enrichissant de nombreux apports, sur la proposition de notre rapporteure, Patricia Demas, qui a effectué un travail Les engagements pris par la filière depuis 2020 pour améliorer la qualité des raccordements à la fibre n'ont pas porté leurs fruits. J'ai moi-même été alerté sur ce sujet la semaine dernière par le syndicat mixte en charge du déploiement de la fibre dans mon département, le Doubs. La qualité et la sécurité des raccordements à la fibre sont loin de s'être améliorées dans la période récente. Il semble même qu'elles se soient dégradées. Cette situation est inacceptable, car elle menace le bon déroulement de la bascule de l'ADSL vers la fibre, qui est désormais bien engagée. Je soutiens donc pleinement cette proposition de loi, en particulier son article 2, qui prévoit de doter les collectivités territoriales de leviers pour contrôler la qualité des raccordements dans les RIP. Cette question me semble essentielle. Alors que la fibre est déployée à partir de fonds publics dans les zones RIP, les collectivités sont souvent démunies face aux dégradations infligées à leur réseau par une sous-traitance peu scrupuleuse. En subordonnant à la qualité effective des travaux le paiement de l'opérateur par la collectivité, cet article

Il s'agit de préciser que l'interdiction du recours au mode Stoc pour la réalisation des raccordements longs et complexes s'applique à la fois aux zones ayant obtenu le statut de zone fibrée et aux communes dans lesquelles la fermeture du réseau cuivre est engagée, ces deux critères étant alternatifs.

notamment à travers la limitation des nouveaux accès au réseau- c'est la fermeture commerciale -, et une phase de fermeture technique pour fermer matériellement le réseau. L'article 3, dans sa rédaction adoptée par la commission, étend l'interdiction du recours au mode Stoc pour la réalisation des raccordements complexes à la fibre aux communes dans lesquelles la fermeture commerciale du réseau cuivre a été engagée. Or, selon l'Arcep, environ 20 millions de lignes étaient déjà fermées commercialement en février 2023. Il apparaît donc plus opportun d'appliquer cette interdiction aux communes dans lesquelles la fermeture technique du réseau cuivre est proche.

plutôt que de viser les communes dans lesquelles la fermeture commerciale du réseau cuivre est proche. Dans la mesure où la fermeture commerciale du réseau cuivre est déjà effective dans de nombreux territoires, cet ajustement me semble pertinent.

est l'avis de la commission ? La rédaction adoptée en commission est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État, qui a consacré l'existence du pouvoir de police spéciale des communications électroniques au profit uniquement du ministre chargé du numérique, de l'Arcep et de l'Agence

électroniques prévoit déjà la possibilité d'une astreinte. En effet, le président de l'Arcep peut demander au président de la section du contentieux d'ordonner à un opérateur de se conformer à ses obligations en cas de manquement susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour le marché.

Cet amendement a deux objets. Tout d'abord, il vise à préciser que le nombre de jours d'interruption du service d'accès à internet est calculé jusqu'au rétablissement de l'accès à internet pendant au moins sept jours, afin de prendre en compte les cas de figure dans lesquels la connexion de l'utilisateur n'est rétablie que momentanément. il tend à clarifier les modalités de remboursement du consommateur lorsque celui-ci a versé des sommes au titre d'une période durant laquelle son service d'accès à internet a été interrompu.

La commission partage pleinement l'objectif de mieux garantir le droit des consommateurs. Cependant, les délais prévus par le dispositif adopté en commission ont recueilli l'approbation de l'ensemble des parties prenantes entendues lors de ses travaux préparatoires. Il me semble donc qu'ils permettent d'assurer un équilibre adéquat entre la protection des consommateurs et la préservation des intérêts économiques des fournisseurs d'accès à internet. Dans la mesure où l'adoption de cet amendement conduirait à remettre en cause cet équilibre, je demande son retrait ; à défaut, l'avis de la commission sera défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Même avis.

cuivre. Dans le cadre de son plan stratégique à l'horizon 2025, la société Orange a annoncé la fermeture progressive de son réseau cuivre au cours de la période 2023-2030. Si cet arrêt est souhaité par les acteurs de la filière, la transition du cuivre vers la fibre doit être assortie des garanties nécessaires pour les usagers, qui se posent un grand nombre de questions. Par ailleurs, le rôle et l'appui des élus locaux dans cette transition vers un nouveau réseau fibre semblent incontournables pour mener à bien cette campagne. Il est essentiel que ceux-ci y soient associés.

et technique du réseau de communication historique cuivre et sur la pertinence du plan d'action retenu pour sa mise en oeuvre. Quel mise en oeuvre. Quel est l'avis de la commission ? . Cet amendement tend à demander la remise d'un rapport sur l'opportunité et les modalités de la fermeture du réseau cuivre d'Orange. S'il ne me semble pas opportun de remettre en cause la fermeture du réseau cuivre à ce stade, dans la mesure où le chantier est déjà engagé, je souscris pleinement aux interrogations des auteurs de l'amendement sur les risques que comporterait un calendrier de fermeture trop rapide et sur la gouvernance choisie pour mettre en oeuvre ce chantier, qui ne permet pas à l'heure actuelle une association suffisante des élus locaux. Cependant, ce texte ne me semble pas être le véhicule approprié pour discuter des modalités de la fermeture du réseau cuivre. Je demande donc le retrait de cet amendement,

est l'avis de la commission ? . Cet amendement vise à rendre l'intitulé de la proposition de loi cohérent avec le champ des dispositifs, qui concernent spécifiquement la qualité des raccordements à la fibre optique et non les enjeux de qualité s'attachant à l'ensemble du réseau. La commission y est donc favorable.

? » Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur, pour une durée de deux minutes ; l'orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute.

Merci

phénomène mondialisé et tentaculaire, aux complicités multiples. Il s'agit d'un braquage des finances publiques. Ce braquage annuel aurait débuté dans les années 2000 pour un montant inconnu, mais sans cesse réévalué.

qui consiste à transférer rapidement et entre plusieurs intervenants la propriété d'actions, de droits ou de titres avec et sans droits à dividendes dans l'objectif d'échapper aux retenues à la source applicables. Lorsque des droits sont attachés à l'action, on parle de Cum ; quand il n'y en a aucun, on parle d'Ex. Il en résulte un double bénéfice frauduleux : non-acquittement de l'impôt et retenue à la source reversée sous forme de crédit d'impôt indûment perçu. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que, depuis 2005, aucune pratique de CumEx n'a été relevée par vos services ? Votre réponse nous intéresse grandement. Mais en tout état de cause, deux phénomènes auraient toujours cours : un phénomène interne et un phénomène externe. Dans le premier, le propriétaire de l'action la prête autour de la date du versement des dividendes à un résident français, le plus souvent un établissement financier. Ce résident français n'est soumis à aucune retenue à la source et rétrocède le dividende à son véritable bénéficiaire, en échange d'une commission. Dans le second cas, l'action est prêtée à un résident dont la convention fiscale avec la France ne prévoit pas de retenue à la source. Ces destinations fiscales sont bien connues, et il faut les nommer : l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Finlande- partenaire européen -, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar. Eh oui ! Je me souviens à cet instant que Jérôme Kerviel avait évoqué ce phénomène lors d'une audition à huis clos, le 8 octobre 2013, dans le cadre de la commission d'enquête sur la fraude fiscale que nous avions conduite, dont Nathalie Goulet faisait partie. Il en décrivait le mécanisme, la pratique connue et reconnue, le gain facile et frauduleux ... Comment croire, dès lors, que l'administration fiscale, avec la compétence qui est la sienne, n'aurait engagé qu'en 2017 des contrôles sur les CumCum dits internes, comme l'affirmait M. Frédéric Iannucci, chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques, devant le Sénat le 1 décembre 2021 Cette administration fiscale, je souhaite la remercier, la féliciter pour sa pugnacité et l'encourager à poursuivre ses investigations sans relâche, à exploiter les documents et les données recueillis dans le cadre des perquisitions engagées, simultanément, dans cinq établissements bancaires BNP Paribas et sa filiale Exane, Société Générale, Natixis et HSBC. Ce coup de filet, conduit par seize magistrats du PNF et plus de cent cinquante enquêteurs, accompagnés de six procureurs du parquet de Cologne, en Allemagne, au titre de la coopération judiciaire européenne, atteste de l'action résolue de l'administration. Ce scandale est d'autant plus choquant qu'il concerne trois des principaux spécialistes en valeurs du trésor (SVT), qui achètent puis traitent la dette française sur les marchés financiers internationaux

S'agissant des sept procédures en cours, je veux préciser que l'une des banques a accepté les redressements, reconnaissant que les pratiques en cause ne relevaient pas du fonctionnement normal des marchés. En revanche, d'autres banques sont dans la dénégation complète ; même face à des cas caricaturaux, avec des prêts de titres la veille de versement d'acomptes, que l'on parvient à démontrer facilement, elles nient le mobile fiscal. » Il y a là de quoi, vous le reconnaîtrez, être optimiste sur l'issue de ces investigations, n'en déplaise au lobby bancaire, qui use et abuse des recours d'obstruction jusqu'à ce que justice soit rendue En effet, la Fédération bancaire française (FBF) a déposé un recours devant le Conseil d'État deux jours après les perquisitions massives. Mais doit-on croire à ce recours ? Il est en effet sans lien avec les perquisitions, mais vise simplement à « mettre un terme à l'incertitude qui existe depuis des années sur le sujet [ ...]. Cela permettra, nous dit le lobby bancaire, à la place de Paris de bénéficier d'un cadre juridique clair, défini par le Conseil d'État et applicable à l'ensemble des acteurs du marché. Nous arrivons au coeur du sujet : le système bancaire tente d'inventer un nouveau concept, aussi innovant que le contournement de l'impôt : la fraude légale ! Le débat pourrait être bref si une quelconque éthique s'immisçait dans les considérations des acteurs de la banque et de la finance internationale. Sur le terrain du droit, comment qualifier une pratique qui a pour seul objectif et pour seule finalité d'échapper à l'impôt ? Quel autre qualificatif que celui de « fraude » doit-on employer ? Le Sénat, le Parlement dans son ensemble et le Gouvernement ne peuvent laisser croire qu'il existerait une forme de fraude légale. Sans attendre l'effort de clarification, feignant d'espérer, la Fédération française bancaire et le Sénat lui-même, par un amendement porté à l'identique

que le ministre du budget, bien aidé par la majorité de l'époque, démonte l'amendement du Sénat et vide de tout contenu notre proposition commune. Il en résulte un dispositif sans substance, sans intérêt et non dissuasif.

Ont été exclues également les opérations de cession, même celles d'apparence frauduleuse, éloignées de plus de quarante-cinq jours ; il suffit donc de nouer son opération de cession le Il ne faut pas, monsieur le ministre, être ingénieur financier pour contrecarrer cette trouvaille législative. M. Iannucci, que j'ai déjà cité, évoquait en ces termes, le 1 décembre 2021, l'efficacité de l'article 119 A du code général des impôts » : « Je répète que nous ne disposons malheureusement pas d'éléments de bilan à ce stade. Je n'ai pas l'impression que les établissements financiers sont très gênés par la période de quarante-cinq jours, mais semblent s'organiser en fonction. loi de finances pour 2022, afin de donner de la vigueur à cet article, mais le Gouvernement n'en voulait toujours pas. Pour que cessent ces fameuses opérations d'arbitrage de dividendes, il faut que le seul arbitre soit l'administration fiscale. Mais comme tout arbitre, elle doit se doter de règles ; c'était l'objet de nos amendements communs.

Notre responsabilité, c'est d'être capables d'identifier cette fraude et de la sanctionner, pour que les fonds dus à la solidarité nationale et à nos politiques publiques soient effectivement versés et recouvrés par l'administration fiscale.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat qui nous est ici proposé intervient dans le contexte d'un scandale de fraude fiscale aggravée, qui aurait coûté, selon les estimations, près de 33 milliards d'euros à l'État français ces dernières années 33 milliards au moment où le Gouvernement fait passer en force et alors que l'urgence est avérée une réforme sociale injuste pour nos concitoyens, visant à combler un déficit de 13,5 milliards d'euros afin de financer d'ici à 2030 notre système de retraites, au moment où nous constatons qu'une proportion significative d'opérations échappe toujours à l'imposition, sans que l'administration fiscale dispose des moyens juridiques suffisants pour y faire échec ... Tragique ironie qui consiste à faire peser sur l'ensemble de nos concitoyens le poids de la dette, alors que l'urgence commande des actions rapides et efficaces contre le détournement fiscal et que la justice fiscale, si précieuse pour le consentement à l'impôt, nécessaire à notre pacte social, nous intime, pour rester une société unie, de préserver notre modèle de solidarité. Ces dernières années ont été marquées par la publication dans la presse d'enquêtes mettant en lumière des systèmes à grande échelle d'opacification de flux financiers- ,, -, financiers- ,, -, illustrant parfaitement le caractère systémique et quasiment industriel de l'évasion fiscale. Ce constat confère aux responsables politiques, quels qu'ils soient, une responsabilité majeure. Si nous ne pouvons nier les efforts réalisés ces dix dernières années et les progrès que représente la création du PNF, de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions

Plus de quatre ans après l'adoption de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, et à la suite de la conduite d'une première enquête sur les pratiques d'arbitrage de dividendes, connues sous le nom de, un consortium de

Cela révèle, malgré les efforts faits ces dix dernières années, l'ampleur du travail qui reste à effectuer et l'urgence que constitue ce problème fondamental pour nos finances publiques, mais aussi pour notre pacte social et démocratique. Je saluerai à ce titre le travail important et régulier que la commission des finances et le Sénat dans son ensemble mènent sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ces dernières années, au gré de la mise en lumière de nouveaux schémas de dissimulation. C'est d'ailleurs précisément à l'issue de ces travaux que notre assemblée avait à plusieurs reprises, et dans le cadre d'un consensus politique, adopté des amendements aux projets de loi de finances visant à faire échec aux opérations d'arbitrage de dividendes. Hélas ! l'Assemblée nationale, en supprimant la partie du dispositif relatif aux montages externes, qui prévoyait un taux de retenue à la source nul pour le versement de dividendes à des résidents étrangers, a altéré l'efficacité de la mesure, qui n'a pu atteindre son plein potentiel, de sorte que ces montages abusifs perdurent. Si nous sommes conscients de la difficulté de la tâche et de la complexité des montages, nous aimerions, car c'est notre devoir, nous assurer que la faiblesse des moyens dont dispose l'administration fiscale face à l'ampleur du problème ne constitue pas une forme de politique. Aussi, monsieur le ministre, nous aimerions connaître les actions que vous entendez rapidement mettre en oeuvre pour pallier les faiblesses juridiques et administratives persistantes, et savoir si c'est avec la même détermination dont le Gouvernement a fait preuve pour conduire la réforme des retraites qu'il mènera de front ce chantier essentiel. Pour conclure, et au nom de mon groupe, je remercie nos collègues d'avoir permis une nouvelle fois d'engager ce débat. Il a le mérite de souligner les efforts colossaux qu'il reste à faire en cette matière : combattre les pratiques délétères destinées à lutter contre cette dimension importante, mais trop négligée, de la crise globale que subit le monde contemporain. La parole

D'abord, sur la question des moyens du contrôle fiscal. Vous le savez, je présenterai prochainement un plan de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières, auquel un certain nombre d'entre vous ont contribué en acceptant de faire partie du groupe de travail que j'ai proposé de constituer à l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le mardi 28 mars 2023 fera date dans l'histoire bancaire française. En effet, des perquisitions ont eu lieu dans pas moins de cinq grandes banques. Cette opération, la plus importante menée par le parquet national financier de toute son histoire, intervient dans le cadre d'enquêtes ouvertes pour fraude fiscale aggravée et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Bien que les investigations soient toujours en cours, ces mises en examen montrent l'importance présumée des fraudes fiscales aux dividendes sur le sol français. En effet, BNP Paribas et la Société Générale, sociétés visées par ces perquisitions, représentent à elles seules 61 millions de clients selon le site Statista. Mes chers collègues, face à un tel séisme, revenons d'abord sur la définition de la fraude aux dividendes. Derrière cette appellation, aux origines diverses et protégées, la manipulation entraînant cette fraude fiscale aux dividendes se nomme le CumCum, une expression qui signifie « arbitrage de dividendes ». Le principe est le suivant : un investisseur non-résident qui détient des actions d'une entreprise cotée en France transfère temporairement, vers la date de versement du dividende, la propriété de ses titres à un établissement bancaire français. Les banques étant domiciliées en France, elles ne sont pas soumises à cet impôt qui concerne les étrangers. L'actionnaire récupère ensuite son titre une fois le dividende versé, mais il faut préciser une chose importante : il est exonéré d'impôt. Par d'ailleurs, nous pouvons mettre le doigt sur un autre phénomène qui constitue qui constitue lui aussi une fraude fiscale aux dividendes : il se nomme le CumEx. Cette pratique a été mise en lumière en octobre 2018 grâce à une enquête menée par un groupe de médias internationaux, intitulée. Le principe de cette opération consiste à à s'échanger, entre investisseurs, la même action autour de la date de paiement du dividende. Cette action entraîne une confusion dans l'administration fiscale qui ne parvient pas à déterminer le véritable bénéficiaire du dividende : chacun reçoit ainsi une attestation fiscale au titre de l'impôt sur les revenus du capital, pourtant payé une seule fois. D'après la même enquête, la fraude aux dividendes aurait coûté au moins 33 milliards d'euros de recettes fiscales à la France entre 2000 et 2020. Nous comprenons donc clairement que les acteurs concernés par cette fraude profitent d'un vide juridique. Le problème étant maintenant identifié, plusieurs questions se posent à nous : quelle réponse législative et/ou réglementaire y apporter, à l'échelle de la France, à l'échelle européenne et internationale ? quel calendrier et avec quels partenaires ? Car, comme toujours dès qu'il s'agit de lutter contre les fraudes, la coopération est une des clés de l'efficacité ! Or, si nous voulons justement gagner en efficacité demain, nous devons bien évidemment trouver des partenaires, qui, jusqu'à présent, n'ont pas souhaité le devenir. Et si nous ne pouvons pas convaincre tous les pays de nous rejoindre dans ce combat contre la fraude aux dividendes, peut-être pourrions-nous les y contraindre encore davantage que ce qui a été fait jusqu'à présent. : comment, concrètement ? Avec quels leviers pouvons-nous établir un rapport de force avec les pays qui, aujourd'hui, sont indéniablement silencieux, voire dans une certaine mesure complices de telles pratiques ? Mes chers collègues, si nous reconnaissons que des réponses à l'échelle européenne ou internationale sont complexes et délicates à mettre en oeuvre, il n'en demeure pas moins que nous pouvons d'ores et déjà apporter une réponse au vide juridique existant au sein de notre droit positif français. Je me rappelle les débats que nous avions eus lors de l'examen des projets de loi de finances en 2019 et en 2022. Je me souviens notamment du dispositif initialement proposé par notre collègue Albéric de Montgolfier, repris par le rapporteur général Jean-François Husson. Les schémas abusifs s'appuient sur des opérations de prêt ou de cession de titres, qui sont des opérations très courantes de couverture de position et font partie de l'activité normale des marchés, en France comme ailleurs. Il convient donc de ne cibler que les situations abusives dans lesquelles le non-résident évite délibérément la retenue à la source sur les dividendes. Sur le plan international, l'instrument multilatéral (Beps), ou érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices, qui a été ratifié en 2018, vient progressivement modifier nos conventions. Dans quelle mesure cet instrument permet-il précisément de remettre en cause les avantages des conventions en cas

plus avantageuse d'un traité bilatéral d'investissement (TBI) signé entre un État dont ils n'ont pas la nationalité et l'État hôte dans lequel ils ont investi. Bien évidemment, je ne suis pas le seul à le penser : j'espère que le plan antifraude que vous présenterez bientôt, monsieur le ministre, permettra de gagner en efficacité pour endiguer ce phénomène mondial. lutter contre les fraudes, c'est agir sur bien d'autres aspects tout aussi importants pour notre démocratie. En luttant contre les fraudes sous toutes leurs formes, nous agissons pour restaurer la confiance de nos concitoyens dans l'action publique. En ces temps où notre administration et nos institutions sont sans cesse remises en cause, tantôt à juste titre, tantôt injustement, je crois, mes chers collègues, qu'un tel combat est crucial. Tellement crucial qu'il doit être l'une de nos boussoles. C'est une priorité pour le Président de la République et, en tant que parlementaire, je poursuivrai mon engagement

est d'être capable d'identifier les bénéficiaires effectifs des flux. Vous avez parlé de la nécessaire coopération avec un certain nombre de pays ; nous

réaliser les démarches permettant d'identifier le bénéficiaire effectif des flux qui sont engagés au titre du versement des dividendes, de la même manière qu'ils ont des responsabilités sur la question du blanchiment par exemple, avec des dispositifs et des clauses qui existent

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au lendemain de la mobilisation de près de deux millions de Français pour demander plus de justice sociale tout en exprimant une très grande hostilité à la réforme des retraites, je salue le choix de nos collègues du groupe communiste d'avoir proposé un débat sur le phénomène mondialisé des fraudes fiscales aux dividendes. Il est de notoriété publique que nombre d'entreprises multinationales utilisent des stratégies de réduction de leur imposition. Ces pratiques représentent une perte de plusieurs milliards d'euros chaque année en recettes fiscales. Cela a des conséquences directes sur les services publics et les politiques sociales essentielles. Les experts évaluent la fraude fiscale globale entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Ce volume nécessite de trouver des solutions, singulièrement en des temps budgétaires difficiles pour nos comptes publics. Nos concitoyens sont très sensibles à ces questions, car ils sont demandeurs d'équité fiscale entre tous. Je veux ici concentrer mon propos sur les scandales financiers révélés par un consortium d'investigation- qui doit en être félicité -, tels les systèmes complexes des ou des CumCum, dont le circuit a très largement facilité la fuite de dividendes à l'étranger, échappant ainsi à toute imposition. Ce type de pratiques interroge sur la frontière entre l'optimisation fiscale et la fraude, qui est parfois difficile à cerner. à cerner. Néanmoins, à partir du moment où la question de cette distinction est posée, il est évident que notre travail est d'adapter la législation et de réprimer les comportements d'évitement fiscal, qui sont moralement et politiquement inacceptables. Notre commission des finances travaille depuis longtemps sur ces questions, ce qui lui a permis de réagir très vite lors de la révélation de l'affaire en 2018. En effet, président de ladite commission à cette date, nous avions déposé durant l'examen du projet de loi de finances pour 2019, avec Albéric de Montgolfier, alors rapporteur général, un amendement qui visait à apporter une solution aux comportements fiscaux douteux. Celui-ci avait été adopté à l'unanimité par le Sénat. Le dispositif tenait en deux points. Un premier visait à contrer les montages dits internes, lorsque des propriétaires d'actions non-résidents prêtent leurs titres au moment du versement des dividendes afin d'échapper à la retenue à la source. Nous avions proposé d'instaurer une retenue au taux forfaitaire de 30 % sur « tous les flux financiers qui correspondent indirectement à la rétrocession d'un dividende à un actionnaire non-résident ». Les banques ainsi taxées pouvaient obtenir le remboursement de cette retenue fiscale seulement si elles étaient en capacité de prouver que l'objet du prêt-emprunt de titres n'était pas fiscal. Le second point visait à lutter contre les schémas d'évasion ou de fraude dits externes, qui voient des propriétaires d'actions les prêter, toujours autour de la date de versement des dividendes, au résident d'un État dont la convention fiscale signée avec la France ne prévoit aucune retenue à la source. C'est notamment le cas des conventions passées avec nombre de pays de la péninsule arabique. Pour contrer de tels dispositifs de contournement de l'impôt difficilement repérables par l'administration fiscale, la solution proposée consistait cette fois à obliger l'établissement payeur- la banque -à appliquer par défaut le taux interne de 30 %. Là encore, le bénéficiaire aurait pu réclamer le remboursement de l'impôt s'il présentait les justificatifs nécessaires. En résumé, nous avions proposé d'inverser la charge de la preuve. Malheureusement, ce bouclier antifraude a été vidé de sa substance par l'Assemblée nationale durant la navette parlementaire. Je le regrette fortement. En effet, en 2018, nos estimations de pertes pour le budget de l'État étaient évaluées à 3 milliards d'euros Dans les délais écoulés, avec notre dispositif, nous aurions dû produire environ 12 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Ces moyens manquent cruellement dans nos caisses, notamment quand on rapproche cette somme du montant du déficit putatif de nos caisses de retraites, celui que le Gouvernement souhaite résorber par la réforme aujourd'hui contestée. Monsieur le ministre, pourquoi, avec le gouvernement de l'époque, n'avez-vous pas soutenu notre amendement ou, à tout le moins, proposé une véritable amélioration du dispositif ? Le Gouvernement s'était engagé en 2019 à nous présenter un bilan de situation pour légiférer de manière pertinente : où en est ce travail ? cette date, aucun nouveau dispositif n'a été élaboré pour véritablement traiter la question que j'évoque ici. Qu'attendez-vous ? Le temps passe, mais le sujet demeure. Aujourd'hui, la prévision de distribution des dividendes des entreprises du CAC 40 est annoncée comme un record pour l'année 2022, celles-ci affichant plus de 140 milliards d'euros de résultat net. En cette période, les Français comprendraient mal s'il devait encore y avoir des dividendes échappant à toute taxation. Concernant les procédures en cours, dont vous avez dit, monsieur le ministre, qu'elles étaient largement médiatisées, il faut distinguer les perquisitions, que j'imagine actionnées par la justice, et une perspective d'accord entre l'administration fiscale et le Crédit Agricole. Est-ce le retour du verrou de Bercy ? Dans tous les cas, il n'est jamais trop tard pour agir. À défaut de meilleurs dispositifs, notre bouclier antifraude reste à la disposition du Gouvernement et pourrait produire rapidement des effets utiles pour nos comptes publics.

que nous venons de parvenir à un accord avec l'administration de la Finlande, qui fait partie des rares pays avec lesquels notre convention fiscale prévoit aujourd'hui un taux nul de retenue à la source,

vous ne serez pas étonnés que je me félicite de ce débat demandé par mon groupe, qui nous permet de prendre un peu de hauteur face à l'amalgame que ne cesse de faire le Gouvernement, en mettant sur un pied d'égalité la fraude fiscale et la fraude dite sociale.

Pour cette seule infraction des CumCum, pour seulement cinq banques, le montant indûment détourné des caisses de l'État pourrait s'élever à 3 milliards d'euros. Trois fois plus que la priorité politique gouvernementale du moment Je vous pose donc la question, monsieur le ministre : disposons-nous bien de tous les outils législatifs pour préserver nos recettes fiscales de la fraude aux dividendes ? Vous avez commencé à y répondre, mais j'aimerais que vous alliez plus loin. Aucune disposition n'a pourtant été prévue dans le dernier budget, si ce n'est de rejeter les propositions quasi unanimes du Sénat pour lutter contre ce pillage fiscal qu'est la fraude aux dividendes. Eh oui ... L'administration s'appuie dans ses investigations sur la notion d'abus de droit et, plus récemment, sur une jurisprudence européenne datant de 2019 2019 relative aux « bénéficiaires effectifs » des exonérations fiscales, ainsi que sur une décision du Conseil d'État allant dans le même sens. Ce changement permet de déterminer, en cas de cession de titres, l'entité qui a un réel intérêt économique dans l'opération. Question : le droit français doit-il s'adapter à ce revirement jurisprudentiel ou, en tout cas, l'accompagner ? Les enquêtes en cours ouvertes et diligentées par le parquet national financier attestent d'un phénomène d'ampleur, qui n'est pas nouveau- il a même une certaine ancienneté. Je me souviens que notre ancien rapporteur général, Albéric de Montgolfier, avait montré que le volume d'opérations de prêt-emprunt de titres était, en 2018, multiplié par huit à la période de détachement de dividendes.

de la fraude aux dividendes s'inscrit dans un contexte qui donne- vous en conviendrez -une acuité toute particulière à cette problématique. Premièrement, quand nous cherchons quelques milliards d'euros pour les retraites, mais que les prélèvements sociaux sur les dividendes échappent au financement de la protection sociale, il est difficile de ne pas y voir au moins une partie de la solution.

a produit dès la première année, en 2018, une explosion de 60 % des dividendes versés aux particuliers, qui se sont élevés cette année-là à 23,2 milliards d'euros. La conséquence, comme l'indiquait France Stratégie, est que la fortune

L'année dernière, la folie se poursuivait. La France est le pays qui a connu la croissance la plus importante du montant de dividendes versés en Europe : 59,8 milliards d'euros, soit une croissance de 4,6 %. Une tendance soutenue par 95 % des entreprises, qui ont maintenu ou augmenté leurs dividendes par rapport à 2021. Autant de valeur qui échappe aux travailleurs, aux investissements et aussi, disons-le, à l'administration fiscale. Records de dividendes, records de rachats d'actions, et, pourtant, les dividendes que l'on ne peut pas frauder sont ceux que l'on n'a pas versés

que la était autofinancée et que la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, du fait du surcroît d'activité économique qu'il a engendré, avait permis des recettes supplémentaires conformes à celles que nous retirions auparavant

2019. Je le redis : si mes prédécesseurs et la majorité à l'Assemblée nationale ont à l'époque revu le dispositif adopté ici, c'est pour qu'il soit conforme aux normes supérieures, à savoir la Constitution et nos conventions fiscales. La réalité, c'est qu'il avait alors été estimé que le risque était trop grand d'une censure totale du dispositif. Celui qui a été adopté a le mérite de pouvoir s'appliquer et d'avoir été validé par le Conseil constitutionnel. Encore une fois, je pense qu'il est trop tôt pour en mesurer les effets

Si nous avons publié un Bofip et si nous n'avons pas proposé une évolution législative, c'est que nous considérons que l'esprit de la loi permet déjà d'aller vers ce que j'ai déjà évoqué : la responsabilité pour les établissements financiers d'identifier le bénéficiaire ultime des flux.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe CRCE nous propose ce soir un sujet épineux, ardu, mais passionnant, et je le remercie, au nom de mon groupe, de nous inviter à cette réflexion. Les membres de la commission des finances se souviennent de l'exceptionnelle audition du 1 décembre 2021 sur les outils de lutte contre les pratiques d'arbitrage de dividendes, au cours de laquelle le chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la DGFiP, M. Iannucci, avait bien du mal à se faire comprendre par le directeur général délégué de la Fédération bancaire française, M. Barel. Entre contrôle de l'encaissement de l'impôt dû et menace de perte de compétitivité des établissements bancaires français à l'échelle mondiale, les logiques se sont combattues avec courtoisie, mais sans concessions. concessions. Tout d'abord, les pratiques en matière de CumCum et de CumEx ont cours depuis maintenant tant d'années que tout se passe, du point de vue des utilisateurs, comme si elles étaient normalisées, voire légalisées. financiers sont désormais tels qu'ils sont considérés comme acquis et que toute tentative de suppression dans un pays rendrait son gouvernement responsable de la perte de compétitivité de ses banques. Dans le même temps, personne ne s'inquiéterait des milliards d'impôts qui échapperaient aux États aux États ... Pourtant, mieux vaut tard que jamais : même si nos administrations fiscales européennes ont eu du mal à appréhender ces phénomènes de fraude, elles méritent tout notre soutien pour ne rien lâcher dans la bagarre et reprendre le dessus. Elles ont surtout besoin de moyens pour parvenir à y voir clair. Comme le dit avec sagesse M. Iannucci : « L'objectif principal est d'identifier les abus, sans toutefois paralyser les marchés financiers, notamment les opérateurs français. » Il ajoute : « C'est un problème de compétences. Comment avoir des vérificateurs suffisamment spécialisés, ayant des compétences pointues sur ces mécanismes ?

Ne pas le faire nous coûtera toujours plus cher : c'est ainsi que l'administration allemande a remboursé plus de dix fois par action la même retenue à la source sans avoir pu vérifier que l'impôt avait été acquitté. Par la mise à jour du Bofip du 15 février 2023 et deux rescrits, notre administration apporte des précisions sur l'application de la retenue à la source aux rétrocessions de dividendes de source française à des non-résidents : elle attaque sous l'angle du bénéficiaire effectif afin de cibler

Oui, il faut traquer les comportements frauduleux, mais sans affaiblir la place de Paris comme place de référence du système bancaire mondial. Oui, il faut agir résolument

en 2018 éclatait le scandale des, révélé par un consortium international de journalistes lanceurs d'alerte. Comme cela a été dit, cette technique d'évasion fiscale frauduleuse consiste, pour les détenteurs d'actions, à détourner la fiscalité sur leurs dividendes.

La pratique des CumCum s'appuie, quant à elle, sur les différences de fiscalité entre pays. Des banques européennes ont ainsi aidé leurs clients à échapper à cette taxe sur les dividendes, avec une perte évaluée, en 2018, à 55 milliards d'euros, pour onze États européens.

En France, il y a un mois, le parquet national financier a conduit la plus vaste opération jamais menée, perquisitionnant cinq banques soupçonnées de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, pour complicité d'évasion fiscale visant à échapper à la taxe sur les dividendes sur leurs actions placées dans des entreprises françaises. Pour mener cette opération, le PNF a mobilisé 16 de ses 19 magistrats,

que je remercie pour l'inscription de ce débat à l'ordre du jour, nous donne l'occasion de rappeler qu'un amendement du Sénat avait été rejeté en 2018 par l'Assemblée nationale et que les recommandations de la mission d'information du Sénat, publiées en 2022, n'ont pas non plus été entendues, malgré des pistes pertinentes comme la production de données sur la fraude fiscale pour le budget de 2024, le doublement du nombre d'officiers fiscaux judiciaires- qui sont 40 aujourd'hui -, la révision des « conventions fiscales internationales prévoyant un taux de retenue à la source nul sur les dividendes », etc. Monsieur le ministre, vous avez mis en place un groupe de travail, dont je suis membre, pour préparer un plan de lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale qui rendra ses conclusions très prochainement. Je ne doute pas que vous tiendrez compte de notre débat. Renforcer Renforcer l'arsenal de l'État, y compris en passant par la loi, est essentiel pour combattre les nouvelles formes de fraude fiscale, avec de nouveaux outils. Il faut aussi des mots justes, et vous les avez employés, monsieur le ministre : ces pratiques sont frauduleuses

En matière de fraude fiscale, le filet antifraude doit être à la fois à fine maille et solide, non pas comme la toile d'araignée, qui, comme chacun le sait, capture les moucherons, mais laisse passer les bourdons.

ce débat, qui s'inscrit dans la continuité des travaux de notre commission des finances et de notre assemblée depuis la publication des en 2018. Dès la divulgation de ces pratiques d'arbitrage de dividendes, qui coûteraient à la France entre 1 et 3 milliards d'euros par an, le groupe de suivi de notre commission des finances sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales s'était immédiatement emparé de ce sujet en proposant notamment un dispositif anti-abus.

Le mécanisme anti-abus a été restreint aux seules opérations de prêt-emprunt de titres, empêchant de mieux lutter contre des montages reposant sur des produits plus complexes. Surtout, l'utilisation abusive des conventions fiscales prévoyant des taux de retenue à la source sur les dividendes de 0 % a perduré, le Gouvernement n'ayant jamais cherché à renégocier ces conventions. Parallèlement, l'administration fiscale, le PNF et les enquêteurs du service d'enquêtes judiciaires des finances et de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ont engagé des travaux pour identifier ces montages

la mission d'information de notre commission des finances sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, dont j'étais le rapporteur, avait salué le travail réalisé par les services d'enquête et appelé à un renforcement de leurs moyens humains. Leur

à tous les montages fiscaux abusifs de grande ampleur, c'est donc d'abord renforcer les moyens des services d'enquêtes et de poursuites. C'est ensuite savoir qualifier ces montages et mettre en place des dispositifs anti-abus véritablement efficaces. Nous savons que le scandale des n'a pas touché tous les pays avec la même ampleur. L'Allemagne aurait subi les pertes les plus importantes, de l'ordre de 50 milliards d'euros. effet, contrairement à la France, le système allemand a permis à certains intermédiaires de demander le remboursement de la retenue à la source sur les dividendes, alors même qu'aucune retenue n'avait été opérée. Ces remboursements indus sont les plus facilement qualifiables de fraude. Les montages, internes et externes, qui se sont développés en France sont plus difficiles à caractériser et se situent à la frontière entre fraude, optimisation et évasion fiscales.

Il convient en effet, pour l'administration fiscale comme pour les enquêteurs, puis les magistrats, de distinguer ce qui relève du fonctionnement normal des marchés de ce qui relève de manoeuvres abusives. Il ne s'agit évidemment pas de paralyser les marchés financiers : le recours à des opérations de prêt-emprunt de titres ou de vente à découvert peut évidemment se justifier d'un point de vue économique, pour assurer la liquidité du marché et pour améliorer le mécanisme de formation des prix. Néanmoins, les autorités de supervision nationales comme européennes considèrent que, si ces opérations sont utiles, elles comportent un risque de déstabilisation et d'abus. L'Autorité européenne des marchés financiers relevait ainsi, en septembre 2020, que les montages internes et externes d'arbitrages de dividendes présentaient plusieurs marqueurs de fraude fiscale. Il faut donc arriver à distinguer ce qui relève du fonctionnement courant des marchés de ce qui relève de l'exceptionnel. Peut-on dire qu'un surplus de valorisation de titres prêtés à la date de détachement de dividendes de 160 milliards d'euros relève du fonctionnement normal des marchés ? cette manoeuvre un objectif avant tout fiscal, pour faire en sorte que les personnes redevables de la retenue à la source sur les dividendes ne soient plus propriétaires du titre au moment de leur versement. Je fais confiance aux enquêtes menées pour nous apporter de premiers éclairages sur la qualification de tels montages d'arbitrages de dividendes. Il nous reviendra ensuite, à nous législateur, d'en tirer les conséquences. Faudra-t-il renforcer le dispositif anti-abus introduit sur l'initiative de notre assemblée ? L'abus de droit et l'identification des bénéficiaires effectifs sont-ils suffisants pour faire toute la lumière sur des schémas potentiellement abusifs ? Comptez sur moi pour poursuivre les travaux de la commission sur le sujet, y compris dans nos fonctions de contrôle. Je rappelle à ce titre que la recommandation n° 20 du rapport de notre mission d'information demandait au Gouvernement de renégocier certaines conventions fiscales pour prévenir la mise en place de montages abusifs. Renforcer les services d'enquêtes spécialisés, évaluer le dispositif anti-abus et renégocier les conventions fiscales : voilà ce que serait une réponse claire au phénomène des. Monsieur le ministre,

qui fait partie de la vie de la société. Les perquisitions menées par le PNF au siège de plusieurs banques en mars dernier feront date. Elles ont remis dans l'actualité deux pratiques financières aux accents latins : les CumCum et les CumEx. Les CumEx avaient déjà fait les gros titres en 2018, lors des révélations de seize médias internationaux, dont. Les perquisitions de mars dernier en sont d'ailleurs la conséquence elles font suite aux enquêtes préliminaires ouvertes en décembre 2021 sur des soupçons de fraude fiscale aggravée et de blanchiment, contre plusieurs grandes banques. Pourtant, ce sont les CumCum qui sont à présent au coeur des débats. C'est sur ces pratiques que le PNF enquête désormais, afin de déterminer s'il s'agit bien de fraude fiscale, c'est-à-dire si l'intention d'échapper à l'impôt est caractérisée. Qu'est-ce qui les différencie ? À peu près la même chose que ce qui différencie l'optimisation fiscale de la fraude fiscale. Dans les deux cas, il s'agit de transférer temporairement un titre financier, afin de diminuer la fiscalité sur les dividendes perçus. Dans les deux cas, le titre est transféré avec le bénéfice du dividende auquel il donne droit. Mais dans le cas des CumEx, la propriété du titre est également transférée afin de tromper l'autorité fiscale. Dans le cas des CumCum, l'opération s'effectue dans un cadre légal, où des intermédiaires opèrent pour le compte des détenteurs de titres afin d'améliorer leur rendement. La première des réponses à la fraude fiscale, c'est la clarification, entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas. Il appartient au Parlement d'écrire la loi et donc de donner cette première réponse. Mais ce n'est pas notre rôle d'entretenir la confusion entre fraude et optimisation fiscales. Cette clarification vaut aussi pour les montants qui sont en jeu. Or, en la matière, le flou prédomine. Comment en serait-il autrement ? Par essence, la fraude fiscale est ce qui échappe au cadre légal, et donc à la calculette de Bercy. Les médias ont diffusé de nombreux chiffres.

la lutte contre la fraude fiscale résorbera notre déficit public ou financera tout notre système de retraite, on va un peu vite en besogne. En tout état de cause, notre groupe soutient une clarification du cadre fiscal applicable aux dividendes. Dans le cas des CumEx, il s'agit de pratiques illégales et de fraude caractérisée. Nous sommes favorables à ce que l'appareil d'investigation et de sanction soit renforcé. Si la France ne semble pas être le pays le plus exposé à ce type de fraude, il est néanmoins nécessaire que nous puissions coopérer au niveau international pour enrayer ces pratiques. Pour les CumCum, le Sénat a été force de proposition dès 2018. Au cours l'examen de la loi de finances pour 2019, plusieurs amendements, dont un de notre groupe, ont été adoptés pour clarifier le cadre existant. Malheureusement, notre proposition n'a pas été retenue par l'Assemblée nationale. Des améliorations ont toutefois été adoptées, comme la contrainte des 45 jours de détention du titre. C'est une avancée notable. Nous proposions à l'époque d'aller encore plus loin, en étendant la retenue à la source de l'impôt à tous les versements équivalant à des dividendes indirects à des non-résidents. Cette solution s'inspire directement du cadre légal applicable aux États-Unis, et plus précisément de la section 871(m) de leur code général des impôts. Elle a l'avantage de réduire drastiquement les dérives, de sécuriser le cadre légal pour les banques et de préserver l'attractivité de la place financière de Paris. J'espère que nous pourrons progresser dans ce sens. C'est ce que les Français attendent de nous. La parole est à M. le ministre délégué.

Éblé, débat qui a lieu deux semaines après que le Gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'une réforme de la lutte contre la fraude fiscale dans notre pays.

le sujet que nos collègues du groupe communiste mettent à l'ordre du jour est important. Monsieur le ministre, vous avez déjà apporté un certain nombre de réponses aux interventions de nos collègues à la tribune, mais pourquoi le Gouvernement a-t-il tant tardé ?

alors que les scandales mondiaux de fraude fiscale se multiplient, révélés par la publication des investigations menées par la presse et par les lanceurs d'alerte, il est urgent d'agir. Heureusement que les révélations des

! Alors que vous avez fait passer une réforme des retraites- vous savez ce que nous en pensons et, surtout, ce que les Français en pensent

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai un peu l'impression d'être dans la chanson de Barbara : « Chaque fois qu'on parle d'amour, [ ...] « C'est avec " jamais " et " toujours ". « On refait le même chemin « En ne se souvenant de rien « Et l'on recommence, soumise, « Florence et Naples, « Naples et Venise. » On parle de nouveau de fraude fiscale ; certes, on en a parlé beaucoup, mais on

Notre collègue Éric Bocquet avait proposé lors d'un énième débat sur la fraude fiscale une « COP fiscale

je suis favorable à ce qu'il y ait une instance indépendante qui permette de placer autour d'une table un certain nombre d'acteurs, y compris des parlementaires et des personnalités qualifiées, pour évaluer plus finement ce que recouvre la fraude dans notre pays. Il est vrai que nous avons des estimations

Madame la présidente, monsieur le ministre, cher Éric Bocquet, mes chers collègues, « tout est dit, et l'on vient trop tard » ... Je vous dirai néanmoins quelques mots sur le sujet important de la fraude fiscale aux dividendes, qui s'est développée au niveau mondial pendant plusieurs années, jusqu'à représenter 140 milliards d'euros- peut-être le casse du siècle Depuis 2018, ces mécanismes d'évitement de l'impôt ont été mis au jour. La plupart des États ont légiféré afin de lutter contre les montages frauduleux, adossés à l'articulation entre législations internes et conventions fiscales internationales. Tout cela est-il suffisant ? Telle est la question qui se pose à nous. Une autre question est celle de l'optimisation fiscale : rime-t-elle avec fraude fiscale ? La frontière entre les deux notions n'est pas toujours simple à tracer. simple à tracer. En effet, nous dit la doctrine, un montage respectueux de la lettre de la loi, mais contraire à son esprit, ne correspond pas à de l'optimisation fiscale et peut être rejeté sur le fondement de l'abus de droit fiscal, sans compter les conséquences pénales éventuelles.

est de constater que les réponses apportées par le législateur sont insuffisantes et que le secteur bancaire, sans violer directement la loi, a profité d'un encadrement trop large de ces pratiques. Sur le fondement, pour être précis, de l'abus de droit, les banques sont actuellement sous le coup de procédures diligentées par le PNF, institution à fort poids politique. Le secteur bancaire, pour prouver sa bonne foi, peut-être par nécessité, a saisi le Conseil d'État. Légiférer à nouveau sur l'encadrement de ces pratiques emporte donc plusieurs conséquences qu'il convient de considérer. D'abord, les marchés financiers et le système bancaire, directement au contact de la mondialisation, ont besoin de sécurité juridique afin de ne pas créer de la crainte chez les investisseurs. Ensuite, bancaires doivent rester compétitifs face à leurs homologues étrangers. Enfin, les banques ont une image dégradée auprès des citoyens, pour qui elles incarnent une puissance capitaliste peu régulée et avide de profits, responsable de crises et affranchie d'une certaine justice fiscale,

bancaires français, leaders sur les marchés européens, doivent être compétitifs, notamment dans le contexte concurrentiel de l'Europe, où ils occupent une place dominante. La pratique du CumEx était connue depuis longtemps par l'administration fiscale, qui faisait visiblement preuve de tolérance. Ensuite, le risque d'interdiction pourrait entraîner un désavantage pour les banques françaises sur la scène internationale, notamment face aux Britanniques depuis le Brexit. Le CumCum profite des failles des conventions fiscales internationales ; la solution pourrait être de modifier nos conventions en ce sens. M. le ministre a rappelé les avancées à ce sujet, notamment au travers du cas de la Finlande. On peut dire aussi qu'une régulation de ces pratiques pourrait être plus efficiente au niveau européen et à l'échelle de l'OCDE.

en matière de contrôle, la DGFiP semble délaisser le fondement de l'abus de droit pour utiliser l'angle du bénéficiaire effectif, qui pourrait être plus efficace juridiquement. À la suite de l'affaire CumEx a été évoquée la possibilité de généraliser les conventions fiscales bilatérales imposant une retenue à la source sur les flux de dividendes sortants. Monsieur le ministre,

sachant que les États-Unis ont mis en place un mécanisme de lutte contre l'arbitrage des dividendes étendu aux produits dérivés. De toute évidence, les CumEx, les CumCum et autres dispositifs de fraude, au regard de leurs répercussions médiatiques très fortes, peuvent sonner le glas de toute possibilité d'optimisation fiscale. Il est donc urgent d'agir, de combler les vides juridiques, comme nous l'avons tous indiqué, et d'avoir une approche éthique de la fiscalité mondialisée si l'on souhaite qu'il y ait encore une acceptabilité de l'impôt, c'est-à-dire, finalement, un consentement à l'impôt. La parole

des informations comme celles qui ont pu être diffusées et relayées par des consortiums de journalistes ou des lanceurs d'alerte, la réponse, à mon sens, est non. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan de lutte contre la fraude fiscale que je présenterai très prochainement, je proposerai que soient mis à la disposition de l'administration fiscale des outils supplémentaires pour aller chercher l'information. Je sais que cela fera débat, qu'il y aura des oppositions, mais, en tout cas, j'assumerai de défendre cette position. Je suis ravi de voir que vous êtes sur la même ligne. Elle peut rassembler très largement

travaillent d'arrache-pied pour identifier les abus et la fraude, sans jamais perdre le sens de la mesure ou du discernement et sans jamais renoncer à faire très précisément la part entre ce qui relève de l'abus et ce qui relève de la bonne foi. Je m'adresse à ces agents afin de les remercier pour leur travail exceptionnel.

tout ce qui a été décrit par l'ensemble des intervenants. Autrement dit, elles nous font perdre des recettes fiscales et gagnent de l'argent avec ces pratiques puisqu'elles perçoivent une commission. En aggravant les pertes fiscales, elles aggravent la dette ; dans le même temps, ces banques sont chargées de gérer nos titres de dette sur les marchés financiers internationaux ! J'ai sous les yeux le code de déontologie de l'Agence France Trésor (AFT) que ces banques s'engagent à respecter. Je cite l'article A.5 : « Le respect par les SVT des règles de bonne conduite et des pratiques professionnelles applicables à leurs activités sur les marchés de taux en Europe est pour l'AFT un élément important de la qualité du service qui lui est fourni.

présente charte, l'AFT peut décider de suspendre le SVT de tout ou partie de ses opérations pour une période qu'elle détermine et abaisse l'appréciation qualitative du classement annuel. Morgan Stanley, avait subi cette sanction administrative en 2020, si vous vous en souvenez, monsieur le ministre : elle avait été suspendue de ses fonctions d'août 2020 à novembre 2020, pour y être ensuite rétablie. Indépendamment